La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance. A été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation.-- y en a-t-il en séance. J'ai bien noté une observation, je vais lui donner immédiatement la parole et je donne la parole à Claude Malhuret où Emmanuel Capus. Pour une mise au point, au sujet d'un vote.-- Merci, monsieur le Président. Je souhaitais effectivement effectué une rectification de vote sur le scrutin, numéro 93, les sénateurs Alain Marc Franck Menonville et Pierre-Jean vers Zlin souhaitaient voter pour. Et le reste du groupe les indépendants souhaitaient s'abstenir.-- Et acte et donner de votre observation le procès verbal est adopté sous les réserves d'usage. Cette observation sera donc incluses. Elle sera inscrite et publié au Journal officiel. Figurera dans l'analyse politique du scrutin concernait. L'ordre du jour. Appelle les explications de vote et le vote à la tribune. Du projet de loi de finances pour 2023. Je vais donner la parole à notre collègue Rémi Serrault pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

la discussion en séance du projet de loi de finances ne nous aura pas pour autant rassurés. Par assuré car les hypothèses même de ce budget sont irréalistes. 1% de croissance alors que personne n'y croit. Pour l'an prochain. Même pas le président de la République désormais si j'en crois ses propos.-- Pas rassuré car l'inflation risque de se poursuivre au-delà de ce que prévoit le gouvernement et a des conséquences immédiates sur la vie des gens et ce sont les meilleurs, les plus précaires qui la subissent de plein fouet.-- Pas rassurés non plus lorsqu'on lit dans la presse que les discussions entre le gouvernement et les républicains sur la loi de programmation des finances publiques ne remettrait rien en cause des dépenses des baisses fiscales prévues mais exercerait un coup de rabot supplémentaire sur les politiques publiques. Dès la première année du quinquennat, le gouvernement nous propose donc un nouveau budget injuste traduisant encore une fois sa volonté de concentrer les baisses d'impôts sur les entreprises et les Français les plus fortunés. C'est un choix que partagent la majorité sénatoriale et que nous ne sommes malheureusement Paris parvenu à rééquilibrer. Vous restez. Dans le même schéma.-- Réduire les ressources de l'État et contraindre ses dépenses votre politique de l'offre est un échec mais vous la poursuivez coûte que coûte. Continuer à dévaloriser les revenus du travail par rapport aux revenus du capital. C'est cela la réalité de la politique fiscale qui est menée, c'est cela la vision de la valeur travail par le gouvernement. Et nous n'auront pas été assez nombreux pour que le sénat adoptent une véritable taxe sur les superprofits de toutes les grandes entreprises ou celui-là ou sur la distribution pardon des super dividende et pourtant.-- La gauche n'aura pas été seul à défendre un peu plus de justice et de redistribution. Je tiens à le saluer.-- Si le Sénat n'aura pas remis de la justice dans ce budget nos travaux n'auront pas été inutile. Néanmoins, car nous avons obtenu des avancées pour les collectivités territoriales. Alors que les finances des collectivités sont mises à mal par l'inflation est menacé par l'explosion des coûts de l'énergie, nous avons obtenu que l'indexation de la DGF sur l'inflation pour 2023 soit votée par le Sénat et nous avons voté l'élargissement du filet de sécurité. Nous avons également adopté la baisse du taux de TVA à 5 5 sur les transports publics. Voilà une baisse de taux de TVA indispensable dans la période. Et nous avons annulé la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée. La fameuse CVAE je rappellerai au gouvernement comme l'a fait notre président de la commission des finances Claude Raynal qu'il revient au Parlement de voter l'impôt. Or ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat ne se seront prononcés pour la suppression de la CVAE. Il faut le noter.-- Enfin malgré leur rejet par l'Assemblée, puis par le Sénat, lors de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques, le gouvernement avait réintroduit dans ce PLF, l'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités par des pactes de confiance qui portent bien mal leur nom et permettent de sanctionner certaines collectivités hier soir. Nous avons à nouveau supprimer à une majorité extrêmement large ce mécanisme coercitif. La question est aujourd'hui posée au gouvernement, Monsieur le Ministre, que restera-t-il de nos votes en faveur des collectivités dans le budget final avec ou sans le rouleau compresseur du 49 3. Êtes-vous prêt à écouter le Sénat quand il porte la voix des territoires au-delà des clivages partisans. Car pour le reste. Si le volet recettes n'est pas satisfaisant, le volet dépenses ne l'est pas davantage. Bien sûr, des efforts sont engagés dans le domaine régalien. Nous avons su le reconnaître mais aurez-vous la capacité de les poursuivre dans la durée. Et sinon nous sommes très loin du compte. Quand on connaît les besoins du pays en matière Southall social dans le domaine éducatif pour la transition écologique. Est-ce que ce budget est à même de relancer la construction de logements à l'évidence non. Est-ce que ce budget répond aux difficultés immenses de l'éducation nationale si peu. Est-ce que ce budget est à la hauteur de la crise écologique dont l'été 2022 aura été l'ultime révélateur. Non. Quelles que soient les discours. Nous en sommes loin. Est-ce que le budget permet de faire face à l'explosion des prix de l'énergie. Rien n'est moins sûr, comme l'ont illustré nos débats dans la nuit de vendredi à samedi. Est-ce que le budget permet de résoudre les difficultés du ferroviaire et le risque d'effondrement des transports publics en Île-de-France. Non et nos débats auront montré que le gouvernement et les amis politiques de madame Pécresse se renvoient la balle sur le dos des usagers. Je pourrais poursuivre sur tant de sujets. Si j'en avais le temps mais je ne veux pas omettre un sujet celui de l'aide médicale d'État, à laquelle s'est attaqué la majorité sénatoriale, y voyant un outil de lutte contre l'immigration. Quand elle ne devrait être considéré que pour ce qu'elle est un outil de santé publique indispensable et qui protège toute notre société. nous autres nous refuserons donc le dogme du moins d'impôts qui bénéficient presque toujours au même, c'est-à-dire les entreprises et les plus riches il contraint le gouvernement à reporter la charge sur l'ensemble des Français et à renoncer à des politiques essentielles. Ces temps-ci. Monsieur le Ministre, que vous préférez. Avec la réforme de l'assurance chômage. Taxer les chômeurs à défaut des super profits avant d'engager une réforme des retraites dont le but avoué est purement comptable. C'est ainsi que nos grands services publics continue à se dégrader l'hôpital l'école, les transports publics la présence de l'État sur les territoires tous nos débats en témoignent. Alors notre vote sera bien sûr négatif. Mais avec l'espoir que sur certains points précis et en particulier pour les collectivités locales. Nos travaux, nos débats nos votes été utile, c'est désormais la responsabilité du gouvernement et de sa majorité relative. Je vous remercie. La parole est maintenant notre collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste avait la parole. C'est le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.-- Je ne doute pas que la citation qui suit vous fera plaisir.-- Je ferai en sorte qu'à l'avenir il soit interdit de financer les dépenses de tous les jours par la dette. Ces mots les doigts. Monsieur Nicolas Sarkozy dans son projet présidentiel de 2007.-- Comment ne pas regarder avec ironie ce budget proposé en déficit à 4,9%, suite au vote de la première partie, soit près de 160 milliards d'euros, excusez du peu. Un besoin d'endettement de 270 milliards d'euros en 2023. À l'heure du retour du principe de souveraineté dans le cadre idéologique de l'exécutif. La dépendance aux marchés financiers demeure plus que jamais.-- La révision constitutionnelle a tendu à sacraliser les lois de programmation des finances publiques qui, sans aller jusqu'à une règle d'or intangible a contribué à réduire le Champ d'expression du Parlement.-- Le droit d'initiative des parlementaires corseté par les règles de recevabilité financière ont une nouvelle fois miné l'examen de ce texte.-- La responsabilité des parlementaires et lorsqu'on examine les dépenses à chaque moment engagé une irresponsabilité matérialisée par l'impossibilité de proposer une dépense 100 piller les crédits d'une autre politique publique. Il ne fait décidément pas être bon pour être progressiste sous la Ve République.-- Le calendrier contraint à déboucher sur des situations a minima ubuesque. Si ça n'était si grave qui ont obligé les parlementaires de tous les bancs a retiré l'intégralité de leurs amendements dans le cadre de la mission Agriculture notamment. Pressé vous mes chers collègues, le 8ème 49.3 doit d'intervenir au plus vite. La démocratie parlementaire on sort abîmée meurtrie du peu d'égards, qui sont manifestés à nos débats. Le projet de budget sort du Sénat comme il est arrivé en matière de taxation du capital.-- Le gouvernement et la majorité sénatoriale se sont rejoints pour refuser ensemble une nouvelle modalité d'imposition des multinationales fondée sur le chiffre d'affaires afin de lutter contre l'évasion fiscale, le rétablissement d'une véritable exit tax pour lutter contre les évadés fiscaux. La taxation des superprofits indispensables mesure de justice fiscale. Un accroissement de la taxe sur les transactions financières, un accroissement de la taxation des dividendes versés un accroissement de la taxation des dividendes reçus. Il ne s'agit pas seulement d'un refus d'impôts supplémentaires. Il s'agit d'un front commun d'une union sacrée contre l'imposition du capital d'un front commun contre la justice fiscale la plus élémentaire. La France c'est une anomalie européenne dans un contexte d'inflation des prix de l'énergie des prix de l'alimentation qui percute nos concitoyens et concitoyennes nos entreprises et nos collectivités. Pourtant, le 28 juillet 2022 quand la président de notre groupe Éliane Assassi interrogé la Première ministre sur le double langage du gouvernement en matière de taxation des superprofits à Matignon souffler de l'air chaud à Bercy on expiré de l'air glacial dans un même temps dans le gouvernement a le secret. Voici la conclusion qu'apporter madame Borne à notre collègue je cite. Madame la présidente. Nous serons attentifs à ce que chacun prenne ses responsabilités et nous serons prêts à agir s'il le faut, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, apparemment il ne l'a pas fallu après une soixantaine d'heures de débat pour la première partie du projet de finance. Nous avons compris que le gouvernement refusait d'entrevoir toute taxation supplémentaire sur le capital.-- Il n'y a pas de versements indus. Le dividende 44,3 milliards pour le second ou le seul second trimestre, ce n'est pas un record, il n'y a pas d'inflation différenciée selon que l'on est aisé ou pas il faut rehausser toutes les tranches du barème de l'impôt sur le revenu pour le gouvernement, il n'y a pas eu de super profits indus. Le gouvernement allant même jusqu'à laisser entendre que l'armateur CMA CGM connaissait une période de difficulté après des profits records. Il n'y a pas de super-profits, à part pour quelques producteurs d'énergie et Total ne réalisent des profits sur son activité pétrolière que sur ses raffineries. Il ne faudrait pas croire, comme on l'entend que les versements de dividendes émane d'une reprise de l'activité économique. Pas du tout il débouche de politique fiscale accommodante favorable incitatives décidées lors du précédent quinquennat.-- À titre d'exemple, en 2018, l'année suivant la mise en place du prélèvement forfaitaire unique la fameuse flat tax. Les dividendes éligibles autant augmenté de 61% à 23,2 milliards d'euros jusqu'en 2020, le niveau était toujours stable, signe que la crise sanitaire n'a pas enrayé la distribution de dividendes. Sans surprise, en tout cas pour nous, un petit nombre de ménages les super-dividendes supérieur à un million d'euros ont eux aussi explosé à 24% des dividendes versés, contre seulement 10% en 2017. Pour rappel, un million d'euros, c'est 90.334 heures de travail au SMIC horaire brut 2580 semaine de travail. 50 ans de labeur. Vous l'aurez compris ce budget pour 2023 est un budget pour rien si peu pour nos compatriotes rien pour l'avenir. Après ça va refuser les propositions de recettes il fallait toute l'inventivité de la majorité sénatoriale et du gouvernement pour expliquer que nos concitoyennes et nos concitoyens. Allez voir la facture d'électricité explosé cette année de 15% après une augmentation de 4% l'année précédente après une envolée de 50% sur les 10 dernières années.-- Les Français payait avant la guerre en Ukraine, les décisions coupable d'ouverture au marché de l'énergie et les sous-investissement chronique dans l'énergie nucléaire. Le bouclier énergie n'y peut rien. Même à 45 milliards d'euros alors que nous aurions pu faire mes chers collègues. Autrement, avec des recettes supplémentaires. Un mot enfin sur les collectivités territoriales. Dans un contexte où les élus ne se mettent même plus en colère, ils se sentent condamnés à subir il bataille dans leur coin ne se révolte pas, mais font beaucoup discrètement au quotidien. Ils attendaient une rallonge du petit filet de sécurité pour 2022 indiscutablement un parfait, même si le Sénat l'améliore c'est toujours insuffisant. Une seule proposition qui va et pour répondre à la préoccupation des élus locaux partout dans tous les territoires. Le retour aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz pour toutes les collectivités. C'est la proposition de notre groupe qui sera débattue ici même demain.-- Quel sort adviendra de ce texte qui sort du Sénat, le Sénat c'est déjà lui-même dédie en faisant voter la suppression d'amendements adoptés s'appliquant à lui-même une forme de 49.3 interne sans grande illusion. Nous le disions en préalable de ce débat sur le budget. Un 8ème 49.3 s'abattra sur l'Assemblée nationale tout en feignant le dialogue le gouvernement aura les coudées franches pour retenir les seuls amendements auxquels elle accordera ses préférences. Nous l'affirmons ici ce serait un casus Belli de revenir sur le maintien de la cotisation sur la valeur ajoutée dans Doris sa suppression la CVAE. Le gouvernement, ça donne un jeu de dupes auquel le Sénat a malheureusement accepté de jouer. Nous le regrettons, nous voterons contre ce budget.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Tout au long de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2023. Notre groupe a eu à coeur de suivre une ligne qui nous semble claire et cohérente. Guidé par de constantes. D'une part. Veiller à contenir notre déficit et notre endettement.-- Bien sûr, en limitant autant que possible les dépenses de l'État mais aussi Arena agissant sur le levier des recettes parce que nous sommes convaincus que nous ne réussirons pas à redresser nos comptes publics sans accroître nos recettes.-- 2ème constante. L'équité fiscale, sociale et territoriale et l'équité. Ce n'est pas à l'égalité de traitement.-- C'est au regard de cette ligne.-- Que nous avons défendu la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits élargie au-delà du seul secteur de l'énergie. Un amendement soutenu par notre collègue Sylvie Vermeillet.-- Cette mesure aurait près permis en 1er lieu. De compenser pour partie les dépenses exceptionnelles que porte ce budget et que nous soutenons par ailleurs pour protéger les Français. Les entreprises, les collectivités face à la hausse des prix, notamment ceux de l'énergie. En second lieu, à un moment où on demande beaucoup aux Français. Comment expliquer que les très très grandes entreprises des plus grandes entreprises qui accumulent des profits records parfois en raison de la crise actuelle ne contribue pas davantage à la solidarité nationale. Ah dépense exceptionnelle, mesures exceptionnelles.-- C'est aussi. Pour ne pas priver l'État de 4 milliards d'euros de recettes cette année et 8 milliards l'année prochaine que nous avons défendu le report de la suppression de la CVAE. Cette suppression. Ne nous paraît pas opportune. Au moment où tant de dépenses sont nécessaires pour faire face à la crise et que de surcroît les données macroéconomiques sur lesquelles est fondée, ce budget sont fragiles, au regard des incertitudes qui pèsent sur le contexte européen et mondial.-- Par ailleurs, nous nous réjouissons que le Sénat nous est suivi sur la presse la suppression de plusieurs niches fiscales un sujet cher à notre collègue Michel Canevet. Dans un double objectif d'efficacité budgétaire et de justice fiscale. Parmi elles. La suppression d'une niche implicite sur la transmission du patrimoine des plus fortunés qui contournent l'impôt sur le revenu en exploitant une faille du dispositif nouveau des PER une anomalie qui coûterait plusieurs milliards d'euros à l'État. Selon certaines estimations.-- Ainsi, plusieurs mesures souvent de justice fiscale. Adoptée par le Sénat en première partie ont permis de réduire notre déficit de 6 9 milliards et sans doute davantage parce qu'un certain nombre de mesures n'ont pu être chiffrés par vos services. Sur le volet budgétaire. Le projet de loi de finances pour 2023 poursuit sa stratégie de hausse des Budgets de plusieurs ministères régaliens. La justice, la santé, l'enseignement, la sécurité, la défense. Nous considérons que ces hausses sont nécessaires pour permettre à ses ministères de mener à bien leur mission qui sont essentiels pour le pays. Concernant les collectivités locales. Sur la DGF notre groupe n'était pas favorable à une réponse uniforme pour toutes les collectivités, parce que nous savons bien que derrière les moyennes parfois flatteuse se cache de fortes disparités aussi. Pour tenir compte de cette réalité et par ces mesures d'équité, nous soutenions le choix d'augmenter la DGF en ciblant les collectivités les plus fragiles. Nous avons eu un long débat Monsieur le Ministre, sur la réforme des critères de répartition de la DSR et des voix se sont élevées sur tous les bancs.-- Pour que le critère de la longueur de voirie communale soit maintenu sa suppression pénaliserait les plus petites communes. Nous comptons sur vous Monsieur le Ministre pour entendre cette voix unanime du Sénat. Concernant la dotation aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménité rural. Le Sénat à renforcer les moyens qui lui sont consacrés pour une meilleure reconnaissance de l'apport de la ruralité à la préservation de notre environnement.-- C'est un message positif adressé aux maires des campagnes de France et nous souhaitons vivement que dans le texte final. Le gouvernement cancer cette belle avancée.-- En matière d'investissements, le nouveau pont vers voter. Doté de 2 milliards d'euros, dont la gestion sera confiée au préfet de département et nous soutenons cette idée viendra compléter utilement la DETR, et la déciles pour soutenir les investissements des collectivités locales. Enfin. Le Sénat a adopté la réintégration des dépenses d'aménagement de terrain dans l'éligibilité au FCTVA. Une mesure, vous le savez très attendu des élus locaux.-- Je veux pour terminer évoquer les mesures visant à protéger les collectivités, les ménages et les entreprises face à l'explosion du coût de l'énergie.-- Nous soutenons le plafonnement de la hausse des tarifs réglementés en faveur des ménages et des petites collectivités.-- Ainsi que l'amortisseur électricité en faveur des collectivités et des entreprises qui nous semble bien ciblés et mieux calibrée à 180 euros le mégawattheure plutôt qu'à 325 comme prévu initialement. Nous voulons saluer cette avancée. Nous avons aussi soutenu l'amendement du gouvernement voté par le Sénat vendredi pour élargir l'éligibilité au bouclier tarifaire Gaz, électricité, notamment en faveur des Ehpads et des résidences autonomie. le Sénat a revu les critères d'éligibilité au filet de sécurité énergie en faveur des collectivités pour le rendre. Plus simple, plus clair, plus efficace. Il nous semble important que vous conserviez au final un dispositif simplifié est suffisamment ouvert.-- Monsieur le Ministre, au terme de ces semaines de débats. Notre groupe d'ailleurs tiens d'abord à vous remercier pour votre présence continue votre écoute.-- Et la facilité de nos échanges. Même si nous aurions souhaité parfois davantage d'ouverture vers les propositions du Sénat. Notre groupe de l'Union centriste à la quasi-unanimité votre rate le projet de budget issues des débats du Sénat.

Ce projet de loi de finances et très inquiétant pour l'avenir car la politique suivie actuellement est une fuite en avant. En matière budgétaire, elle nous conduit dans le mur et nous risquons de nous retrouver dans la situation de la Grèce.-- Une réflexion d'ensemble est en particulier nécessaires sur les conséquences de la politique du quoi qu'il en coûte et sur les séquelles pour la France du blocus économique imposé contre la Russie.-- Tout d'abord la politique du quoi qu'il en coûte. Eh bien cette politique conduit à un endettement massif, en faisant croire qu'on peut toujours continuer à dépenser sans se soucier des conséquences pour l'avenir. Cependant, il n'y a pas d'argent magique. Or depuis le président Sarkozy inclus. Tous nos dirigeants se comportent comme la cigale de la fable et il ne faut pas s'étonner si notre situation France financière et beaucoup plus dégradée que celle de l'Allemagne. Il est vraiment temps de dire à nos concitoyens la vérité à ce sujet.-- Par ailleurs.-- La guerre en Ukraine ou plutôt la décision cautionné par la France d'organiser un blocus économique contre la Russie est une autre source de difficultés. Ce blocus économique a en effet des conséquences très graves pour notre économie.-- Probablement plus grave pour nous que pour la Russie, ce qui est vraiment un coup.-- sur une, sur une grande radio nationale 2 économistes ont ainsi confirmé que le seul boycott du gaz et du pétrole russe. Sans compter le reste. Est à l'origine de plus de 50% de l'inflation.-- Là aussi nos concitoyens qui sont victimes d'une hausse galopante des prix doivent être informés et conscients de cette réalité. Voilà. Monsieur le Ministre, chers collègues. Voilà les raisons pour lesquelles je voterai contre le projet de budget pour 19 La parole est maintenant président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. La parole monsieur le président.-- Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Après une première partie du budget sensiblement augmenté avec la réforme de la loi organique relative aux lois de finances

Comment avait dit lors de la discussion générale, le 17 novembre, le Sénat a délibéré. Une délibération parfois contrainte par les nouvelles règles de l'examen d'. En temps programmé des règles et si on était dans l'ensemble, à l'invitation du président de la commission des finances. Par mois ça ça. Que va-t-il subsister de nombreuses modifications adoptées après cette première lecture alors que la réunion de la commission mixte paritaire a été avancée à ce soir. Et que selon toute probabilité on se dirige, de nouveau, vers un nouveau 49.3 à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous regarderons avec intérêt à la situation actuelle est inédite. Par les deux par les pour les 2 lois de finances rectificative. Cette année l'Assemblée et le Sénat ont su trouver des terrains d'entente. Évitant ainsi de repartir pour de nouvelles lecture. Ne pourrait-on pas en être ainsi pour le PS. J'appelle ça la fait à la modération des uns et des autres, afin de préserver la crédibilité à terme de nos institutions. Les amendements proposés par le gouvernement et adopté par le sénat ont de fortes chances de perdurer. Suppression de la condition d'âge de décès de l'époux, ancien combattant pour la demi-part de sa veuve modalités d'indexation de la déduction pourrait pas précaution. Justement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des énergéticiens ainsi qu'à certain nombre d'ouvertures de crédits dans les domaines de la sécurité civile

aux crédits de la mission Écologie et a le bouclier tarifaire à l'habitat collectif et réévaluation des charges du siège public de l'énergie. Le rejet par la majorité sénatoriale de quatre missions en particulier la cohésion des territoires et l'agriculture n'est pas très surprenant. Il y en a tous les ans et il nous amène à voter sur un budget amputé de nombreux crédits même si la question des missions de l'État dans certains domaines peut légitimement légitimement se poser. Surtout avec le défi encore massif que nous nous apprêtons à souscrire, en 2023, ce déficit pourrait être aggravée par dizaines prévu de la situation internationale. Des prévisions de croissance du gouvernement reste crédible. Bien que la prévision dans ce domaine s'apparente souvent à de la météorologie. La réforme phare de la première partie était la suppression sur 2 ans de la contribution sur la valeur ajoutée, la fameuse CVAE. La majorité sénatoriale a tenté une solution médiane prêt à revoir à la voie la compétitivité de l'entreprise et les finances des collectivités avec un coût budgétaire non négligeable pour l'État mais la CVAE a survécu, du moins au Sénat.

D'abord pour le ciné ça des rayons bientôt souligner départements et de façon massive aujourd'hui pour celui de la sécurité sociale en période d'inflation des prix à la consommation. Cette évolution n'est pas défavorable aux finances publiques. Même si le consommateur en paie concrètement la facture. Le rapport de la Cour des comptes. Cet Automne sur la situation des finances locales étaient éclairant. Au regard des comparaisons internationales. Les finances des collectivités locales. Ne représente un froid que 20% environ de la dépense publique derrière les dépenses de la Sécurité sociale et celle de l'État c'est bien hier à la moyenne européenne où les dépenses des collectivités locales représentent en moyenne 40% de la dépense publique. Il est vrai que le niveau global des dépenses publiques en France reste n'est plus élevé de l'OCDE. En 2023, toutes les missions de l'État ou presque verront leur budget augmenter c'est les c'est d'une part de l'inflation, d'autre part la volonté du gouvernement d'assurer un certain nombres de missions essentielles mais aussi du grand retour du service de la dette avec la remontée des taux d'emprunt. Plus de 52 milliards, 50 milliards

La suppression du critère de potentiel financier pour la dotation du local. Et sur ses de partie le financement des charges débroussailler môme pour les communes à fort linéaire. La majoration de la dotation biodiversité à hauteur de 4 millions ou encore la NT1 intégration du critère de voirie pour le calcul de la DSR. Nous regrettons malgré tout que nombre d'autres propositions n'aient pas été. J'ai pas rencontré le succès, en particulier dans le développement local et durable. Le secteur médico-social et où le secteur patrimonial et culturel sur attaque Jérôme. La suppression de la réforme de la répartition au sein du bloc communal voté l'an dernier nous paraît préférable dans la mesure où la répartition des charges d'aménagement varie beaucoup en fonction de chaque territoire. La répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l'IFER reste assuré complexe qui mériterait davantage de débats. Elle doit en tout cas veiller à rester incitative pour les les acteurs locaux pour l'acceptation de l'implantation des parcs éolien ou solaire. Il nous ôter du PLF 2023 et la possibilité d'amender. Sur les indicateurs du performance et plus largement sur les plafonds d'emplois de l'État et des opérateurs. Nous verrons là, s'il s'agit bien de l'oeil et d'amélioration de l'action publique ou d'un gadget de plus. après ces différentes de remarques et au vu des nombreux points évoqués. Les membres du groupe RDSE. Voteront majoritairement pour l'adoption de ce PLFR 2023 avec néanmoins diversité et liberté de vote oblige quelques abstentions. Merci. Monsieur le président. La parole est à notre collègue Jérôme Bascher. Pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Tout d'abord, c'est le 1er projet de loi de finances que nous examinons avec. La nouvelle loi organique sur les lois de finances que le président rénale s'est. Attelé à bien faire respecter et rien que pour cela pour avoir tenu les aussi les délais dans ce. Nouveau temps contraint, il faut le remercier mais je remercierai d'abord le rapporteur général qui nous aura permis avec vous Monsieur le Ministre d'avoir un dialogue.-- Une contribution, une présence.-- Vous aurez compris. En creux de qui nous notons l'absence ce budget, c'est le budget de la volatilité de la variabilité de l'instabilité. Et de l'inflation.-- Tout d'abord.

Monsieur le Ministre vous avez maintenu cette. Ce point sur les nouveaux ou les anciens contrats de Cahors de lourdes. On a eu tous les termes qui sont apparus. Mais ce qui est certain c'est que la première ministre, vous avez dit le contraire à l'Association des maires de France et nous étions nombreux aux côtés de nos élus locaux. Eh bien ces avis un peu fluctuant ne facilite pas le débat à un moment où on aurait besoin d'un CAP d'un cap politique la. De politique économique d'un cap politique tout court. Alors Monsieur le Ministre, vous avez eu aussi de l'inflation, l'inflation dans les amendements, mes chers collègues, nous sommes passés en 10 ans de 500 à 3000 amendements sur cette loi de finances. Pourquoi pas. C'est le droit du Parlement et nous l'avons utilisé à plein après que l'Assemblée nationale. On a eu été largement privée.-- C'est aussi l'inflation dans la hauteur et les milliards des amendements.-- Un amendement du gouvernement fait plus de 25 milliards et donc un sous-amendement a fait près de 6 milliards. Nous n'avons jamais vu de tels mouvements sur des amendements. Donc il faut peut être retrouvé par. Du du calme là dessus pour bien légiférer trop d'instabilité.-- Enfin. On a eu aussi de la stabilité sur l'article d'équilibre étant donné. Ce qui s'est passé, on s'est trompé de quelle d'un chiffre moins d'un chiffre plus c'est sûr que ce ne sont que des milliards d'euros. Alors à la fin sur l'article d'équilibre, nous obtenons effectivement à déséquilibrer le budget que.-- Nous allons voter très largement dans le groupe Les Républicains n'est pas un budget complet, nous en avons bien conscience, Monsieur le Ministre, c'est aussi la limite de l'article 40 qui ne nous permet pas de reconstruire totalement un budget. Mes chers collègues, nous le savons. Nous vous faisons des propositions car on ne peut pas continuer d'avoir un budget en déséquilibre. 500 milliards de budget, 156 milliards de déficit, 270 milliards.-- D'emprunt de long terme à faire 270 milliards pour 500 milliards de budget l'année dernière, je vous disais qu'on était à la moitié du budget financé par la dette. Nous sommes dorénavant au-delà de la moitié.-- Alors évidemment ça ne peut pas continuer comme cela pour un quart d'un côté vous nous proposez la baisse des impôts et nous pouvons y souscrire sur la CVAE. Nous nous dans le groupe. Les Républicains, nous sommes pour la suppression de la CVAE. Mais pas comme cela, ce n'est ni je ne se fait ni à faire, c'est de l'improvisation comme vous avez improvisé sur la redevance et vous nous avez toujours pas proposé de régime pour remplacer en 2024 ce ce qui est ce qui doit être sur la CVAE. C'est la même chose. Votre mécanisme de compensation aux collectivités locales ne convient pas de convient pas.-- Alors c'est au travail que nous vous appelons et un travail de concertation avant de prendre des mesures comme ça à l'emporte-pièce sur des milliards qui concerne les collectivités.-- Et la compétitivité de la France. Nous vous avons fait des propositions pour reprendre l'invitation du FMI mais aussi ce que le Sénat a voté. Lors de la loi de programmation des finances publiques. Nous vous avons réorienté nous avons diminué les dépenses. Nous y étions engagés dans la loi de programmation en cohérence. Nous avons diminué les dépenses et à la fin, nous réduisons aussi le déficit public, hormis l'émission que nous avons.-- Refuser et pourquoi avons-nous refuser certaines missions, mes chers collègues, ce n'est pas comme ça des tocade que nous aurions.-- C'est que ce sont des secteurs pour lesquels ce ne sont pas les crédits qui manque, c'est la réforme, c'est le courage.-- Absence de réforme sur l'immigration et c'est pour cela que nous avons rejeté les crédits notre agriculture est dans une très mauvaise passe et ici les deux. Les rapports sont nombreux pour le souligner nos alertes sont récurrentes et là encore nous avons refusé les crédits. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin d'argent pour notre agriculture pour la moderniser. Pour. La rendre plus bio plus écologique. Ce n'est pas ça le sujet c'est que vous ne travaillez pas à la réforme et lorsque vous vous ont par exemple des propositions très bien venu comme celle de Christine Avart pour éviter 500 millions d'euros de dépenses pour acheter des voitures chinoises on améliore à la fois le déficit public et à la fois le déficit commercial, voilà le double bénéfice que nous vous proposons. Alors Monsieur le Ministre, avant de terminer, je voudrais quand même car il y aura un 49.3 n'ici eux l'ignorent. Nous ne sommes pas des Garennes de 6 semaines. Il faut retenir quelques points d'attention, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Évidemment il y a la dotation globale de fonctionnement. Évidemment il y a le filet de sécurité telle que proposée par le Sénat qui a reçu l'aval de l'AMF de l'ADF et de l'ARF territoires les territoires réunis, ils ont donné leur aval. Il y a aussi et nous avons alerté très fort et les entreprises continuent de travailler avec vous, je le sais je vous sais attentifs, Monsieur le Ministre là-dessus au mécanisme de contribution de la rente Afra marginal des installations électriques notamment avec des tarifs revalorisés chez nous 145 euros. Du MWh pour le biogaz. Ça doit être cela. Oui ça. Je ne veux pas me tromper sur les. Et puis. Également.-- Nous avons alerté sur la TGAP, si nous avons gelé la TGAP c'est qu'en période d'inflation augmenter aussi la TGAP, le risque c'est les failli les jaunes taxe carbone plus pris de. des carburants, c'est la même chose pour l'électricité, enfin il y a le FCTVA sur lesquels nous y sommes très attachés et dans la dernière ligne droite qui me reste, penser à la TVA pour les chevaux.-- Merci beaucoup.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la commission des finances. Monsieur le rapporteur général. Mes chers collègues.-- Après 3 semaines de débats, de jour comme de nuit, 26, débat sur les missions et les comptes spéciaux et plus de 2500 amendements examinés. Nous achevons l'examen du 1er budget de ce nouveau quinquennat aujourd'hui.-- Et puisque ces moments sont partagés, je tiens tout d'abord à remercier au nom de mon groupe les indépendants. La commission des finances et le gouvernement pour l'engagement pour leur engagement. Cet engagement qui a permis la bonne tenue des débats et la qualité de notre travail.-- Cela vaut particulièrement pour vous monsieur le ministre des Comptes publics. Et pour vous monsieur le rapporteur général. Vous avez passé ici de longues heures et vous avez toujours pris le plus grand soin pour répondre à nos questions et à nos interpellations. Cela améliore grandement la qualité de nos débats. Je tiens également à remercier le président de la commission des finances qui n'a pas ménagé son temps. Mais qui a su ménager le nôtre. La progression. En invitant régulièrement nos collègues les plus prolixes à davantage de concision. Nos débats ont été riches lors de la deuxième partie comme il l'avait été, lors de la première. Nous avons pu débattent de sujets importants pour les collectivités locales et pour les élus.-- Je pense notamment à la mise en place du fond Vert. C'est tout. Il sera à la disposition des acteurs de terrain. Il permettra de faire avancer la transition écologique par des actes, plutôt que par des polémiques. C'est ça l'écologie du réel. C'est ça l'écologie de l'action.-- Nous avons également renforcer les dispositifs pour aider les collectivités à faire face à l'inflation.-- Aujourd'hui le coût de l'énergie. C'est l'angoisse majeure des élus locaux. Ils savent pouvoir compter sur l'état mais ils attendent maintenant les actes.-- Je ne reviens pas sur les dispositifs votés en première partie, notamment le filet de sécurité dont les conditions d'éligibilité ont été supprimé l'indexation de la DGF sur l'inflation. Ces mesures répondait aux inquiétudes des collectivités. Mais comme je l'ai déjà dit à la fin de la première partie, ces mesures ne sont pas ciblés sur les collectivités qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi notre groupe a déposé plusieurs amendements visant à encadrer ces dispositifs non pas pour pénaliser certaines collectivités mais bien pour soulager les finances publiques dans leur ensemble. d'esprit dans ce même état d'esprit que nous avons abordé l'article 40 quater il réintroduise est dans le PLF, l'article 23 de la loi de programmation des finances publiques en instaurant des contrats de confiance nouvelle version adoucie des contrats de Cahors. Ces accords et vise à maîtriser l'évolution des dépenses locales et à renforcer le crédit de la France.-- Ce n'est pas rien.-- Notre groupe avait toutefois exprimé clairement au moment du projet de loi de programmation ses réserves vis-à-vis de mécanisme contraignant. Ces réserves persistent, notamment à cause des sanctions qui sont trop sévères pour les collectivités.-- Mais nous pensons plus opportun d'améliorer les solutions proposées par le gouvernement, plutôt que de les rejeter en bloc. Nous avons proposé de conserver le mécanisme de suivi des dépenses tout en supprimant les pénalités associés. Nous aurions ainsi préféré que le Sénat puisse aboutir à un mécanisme de contrôle des finances locales sans mesures coercitives car c'est là que le bât blesse.-- C'est ce que nous souhaitons.-- J'espère que dans le cadre de la navette. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Cet accord aboutira sur ce sujet qui concerne à la fois les collectivités et nos finances publiques.-- À ce propos, je me réjouis que notre assemblée et puis réduire le déficit public de 0 2 point de PIB.-- Certes, c'est moins que l'objectif que le Sénat s'était fixé en loi de programmation. Mais c'est une avancée probante que notre groupe salue. D'ailleurs, la réduction des déficits et formellement bien supérieur à 0 2 point de PIB. Mais cette hausse est en trompe-l'oeil.-- Car le budget sur lequel nous devons nous prononcer être amputé de certaines missions.-- Et non des mois.-- Or cette carence brouille le message politique que nous envoyons.-- Quel est le message envoyé à nos agriculteurs qui comptent sur notre soutien lorsque le Sénat ne votent pas les crédits de la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales. Quel est le message envoyé à nos élus locaux qui compte aussi sur notre soutien lorsque le Sénat ne votent pas les crédits de la mission cohésion des territoires.-- Quel est enfin le message envoyé à tous nos compatriotes qui souhaite que notre politique migratoire, soit à la fois plus juste et plus ferme. Lorsque le Sénat ne votent pas les crédits de la mission Immigration, asile et intégration. Rejeté ses missions c'est convenir qu'il y a un problème. Certes. Je l'entends bien, mais cela ne dit rien de la solution souhaitée. Cela ne dit pas ce que nous voulons. Mais juste ce que nous ne voulons pas. En conséquence, le texte ne nous paraît pas parfaitement équilibré à ce stade c'est pourquoi. Notre groupe s'abstiendra majoritairement et que certains le voteront pour. Pour conclure, mes chers collègues. Messieurs les ministres, enfin pardon monsieur le Ministre.-- Je voudrais dire un mot des communes nouvelles. À l'initiative de notre collègue que j'entends, Françoise Gatel. Le Sénat a envoyé un message clair.-- Il faut de toute urgence pallier la baisse de dotations qui menacent, certaines communes nouvelles. Le dispositif retenu par le Sénat et peut être améliorer techniquement. C'est pas. Mais j'espère que nous parviendrons à une solution de compromis qui répondra aux attentes des élus locaux. Je pense notamment, mes chers collègues, si vous me permettez aux communes de Douai en Anjou et de Segré en Anjou. Pour elle, il y a une urgence absolue, la situation n'est absolument pas tenable. Mais je pense évidemment. Aux quelques autres communes qui sont concernées. Je vous remercie. remercie. La parole est à notre collègue Daniel Breuiller pour le groupe écologiste solidarité et Thierry. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur général, chers collègues. D'abord après 2600 amendements des dizaines d'heures de débat. Je voudrais vous dire monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur général. Merci pour ce moment. Ce projet de loi de finances procède de choix qui ne nous conviennent pas d'inspiration libérale baissant l'impôt des entreprises refusant toute nouvelle contribution de ceux qui accumulent richesse des dividendes et donnant moins à ceux qui ont peu il accentuera un peu plus les inégalités et les écarts sans cesse plus grand des revenus de notre pays.-- Selon l'Insee, les mesures sociales et fiscales intervenues en 2020 et 2021, profite surtout à la moitié la plus aisée de la population. Elles induisent une augmentation du niveau de vie allant jusqu'à 470 euros annuels en moyenne pour les personnes entre les 7ème et 8ème décile contre 90 euros pour les 50% les plus modestes.-- L'inflation actuelle accentuera encore cette réalité brutale car elle pénalise bien plus les catégories modestes et moyennes.-- La suppression de la CVAE, privant l'État de 8 milliards de recettes en pleine période de crise serait immanquablement répercuté sur les ménages via la TVA ou via l'endettement et contribuerait ainsi à l'affaiblissement du service public. Le bien commun de ceux qui n'ont pas de Patrimoine. C'est pourquoi nous nous y sommes opposés.-- Notre philosophie notre projet politique, celui de la sobriété est structuré sur une qualité de vie garantie pour tous. Et par le fait de demander plus d'efforts à ceux qui accumulent toujours plus plus de richesses plus de bien plus de dividendes et bien sûr qui pollue également plus.-- Si l'immense majorité de nos amendement a été rejeté par la majorité sénatoriale.-- Notre groupe a tout de même tenté d'exposer les termes possible d'un avenir socialement plus juste désirable et durable sur la mission enseignement scolaire qui concerne 12 millions d'élèves, nous avons voté la hausse indispensable de 3 7 milliards de crédits mais la crise et d'une profondeur bien au-delà du simple sujet budgétaires.-- Le budget de la mission économique traduit une politique très généreuse d'aide non conditionnée trop fortement voir essentiellement destinée aux grands groupes et sans en faire un outil efficace de la bifurcation écologique comme si essaye les USA. La hausse des crédits de la justice que nous avons approuvé pour indispensable elle elle ne suffira pas à remettre à flot un système à bout de souffle. Sur le volet sécurité civile notre déception est grande. Les moyens ne sont pas à la hauteur car les conséquences du dérèglement climatique sont et seront chaque année plus grave.-- Des crédits de la mission santé ne suffiront pas. L'hôpital public s'effondre, les déserts médicaux s'étendent nombres de Français renoncent aux soins, la santé mentale est au projet de loi de finances, ce que la psychiatrie est à la médecine un parent pauvre et délaissée il faudrait pourtant aider les adolescents nombreux en souffrance psychique, leur souffrance et celle de leur famille sont si grandes.-- Ce projet de loi de finances n'a pas non plus assez pris la mesure de la détresse de nombreux étudiants. Nous avons proposé plus de justice sociale pour les bourses insuffisante rejeté rejeter aussi toutes les mesures pour le logement pour permettre aux jeunes de se loger et de vivre au pays, malgré la multiplication des airs Bien. Des résidences secondaires et l'envolée de la spéculation immobilière. Rejeter aussi les aides aux autorités organisatrices de mobilité partout en France, alors que d'autres pays européens s'y engouffre réellement. Comment peut-on consacrer des milliards aux déplacements automobiles et simultanément refusé d'aider les transports en commun. La TVA à 5 5. Monsieur le Ministre sera-t-elle maintenue. Nous avons défendu l'augmentation du versement mobilité augmentation qui avait été demandé par Valérie Pécresse pour l'Île-de-France mais refusée par la majorité sénatoriale, la désorganisation des transports va coûter cher cher à la planète en pollution cher aux usagers d'abord mais cher aussi aux entreprises, car les salariés ne pourront assumer leurs horaires de travail avec un système totalement désorganisé. Le gouvernement a fait la sourde oreille durant tous nos débats faire payer 90 euros aux usagers d'Île-de-France, alors que les conditions de transport sont épouvantables et se dégrade encore. C'est inacceptable. Dans le Champ culturel, l'avenir de l'audiovisuel public reste incertain et les menaces qu'au nom de la sécurité des Jeux Olympiques vous faites peser sur la saison 2024 inquiète un secteur culturel déjà fortement fragilisé. Malgré un effort budgétaire réel. Nous craignons des baisses des Budgets locaux pour la culture, qui réalise 9, 8 milliards d'euros d'investissement des trois quarts de l'investissement public. Si les collectivités se trouve face à ces choix, ce n'est pas de gaieté de coeur. Cette loi de finances pourraient grâce aux amendements sénatoriaux préserver un peu leur capacité à agir avec l'indexation de la DGF et un bouclier énergie simplifiée étendue mais respecterez-vous ses choix avec l'article 44. Vous avez choisi de passer au-dessus de tous les votes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cela témoigne d'une défiance à l'encontre des collectivités et du Parlement. Les collectivités ont besoin de confiance, pas de contrat. Enfin d'un point de vue environnemental. Nous sommes loin, très loin du compte. Il aurait été possible de faire au fond le même effort que vous feat pour le bouclier carburant ou mieux encore celui fait face au Covid. Car la crise est d'une ampleur similaire au lendemain de la COP27 à la veille de la COB biodiversité la continuité budgétaire à peine améliorée est un contresens historique, le report à plus tard d'une véritables rénovation thermique pénalisera de nombreux foyers nos émissions de CO2 et notre balance commerciale par la dépendance aux fossiles la défense des écosystèmes la biodiversité la forêt la préservation de la ressource en eau. L'adaptation de notre agriculture vers l'agroécologie. Doivent être érigée en grande cause nationale, c'est une nécessité pour nous, pour nos enfants et pour nos petits enfants enfin ce budget est rendu insincère par le choix de la majorité sénatoriale de supprimer des missions entière plus d'APL plus de passeport de carte d'identité plus d'aides aux agriculteurs plus d'hébergement d'urgence plus de politique migratoire pour afficher une baisse de la dépense publique. Vous laisserez donc le gouvernement décide. Pour Pour notre part, nous ne voterons pas ce budget qui privilégie les baisses d'impôts aux urgences sociales, écologiques et dont par ailleurs toute votre communication, Monsieur le Ministre nous annonce votre choix de le 49.3 Izé dès la semaine prochaine.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Il y a un an une motion tendant à opposer la question préalable avait été adopté, excluant ainsi tout débat sur les différentes missions budgétaires du PLF pour 2022. Notre assemblée était alors privé des nocturnes budgétaire hivernale. Certains en sont peut être nostalgique, vu le dépassement des records d'amendements discutés cette année que ce soit en première partie avec 1741 amendements discutés ou en seconde partie. Mes chers collègues, ce projet de loi de finances pour 2023 a été l'occasion d'adopter des mesures positives pour notre pays pour les ménages, les services publics et les collectivités. À commencer par le pouvoir d'achat des ménages avec l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, qui représente 6,2 milliards d'euros. Un budget au service de nos missions régaliennes également avec des efforts considérables pour le ministère de la justice. Un budget en augmentation de 8% pour la 3ème année consécutive. Pour le ministère de l'Éducation nationale aussi avec la revalorisation des salaires des enseignants. L'objectif étant le salaire minimum de 2000 euros nets par mois en début de carrière. Un budget à l'écoute des collectivités enfin avec l'augmentation en 2023 de la dotation globale de fonctionnement de 320 millions d'euros. Après des années de baisse, le maire que j'ai été entre 2001 et 2017 s'en souvient douloureusement moins 14 milliards d'euros, puis de stabilisation entre 2017 et 2022 la DGF augmente pour la première fois depuis 13 ans et je veux encore. Une fois encore la rappeler en cette période si délicate pour les collectivités locales.-- Cependant force est de constater qu'à l'issue de son examen au Sénat. Le projet de loi de finances pour 2023 et dénaturé. Raison pour laquelle le groupe RDPI s'abstiendra sur l'ensemble du texte en cohérence avec notre position d'abstention sur la première partie du texte en réalité dès l'examen de cette première partie les fondations de ce budget pour 2023, été défiguré. Les amendements adoptés sur l'indexation de la DGF et sur le fil le filet de sécurité. Ils sont pour quelque chose mais la suppression ubuesque de la réforme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises enfonce définitivement le clou. Idée de dégrèvement improvisé pour justifier votre report, après les sénatoriales entre les réunions de commission et l'examen du texte en séance. Oui, ubuesque rejet des amendements de suppression de la réforme de la CVAE puis dégrèvement improvisé pour ensuite rejeté l'article que vous aviez pourtant modifié. Le gouvernement veut proposer de supprimer la CVAE, mesure qui bénéficierait à 530.000 entreprises dont 25% des gains seraient fléchés vers l'industrie. Chers collègues, je m'interrogeais déjà sur la cohérence de la majorité sénatoriale en cette fin de période où tu automnal. Tout en saluant la courtoisie et l'écoute de notre de notre rapporteur général. Je constate que mes, mes demandes sont visiblement restées lettre morte. Dénaturé sous le chaud en première partie, le projet de loi de finances l'est tout autant. D'un point de vue budgétaire en 2ème partie, arrêtons-nous un instant sur le bilan de l'examen d'émission agriculture cohésion des territoires, immigration, Immigration, asile et intégration administration générale et territoriale de l'État et on l'a vu hier soir aussi lors de l'examen de la mission Aide publique au développement, avec un amendement de suppression de 200 millions d'euros les crédits de ses missions pourtant primordial dans l'ossature budgétaires ont été. Résultat, 33,7 milliards d'économies en trompe-l'oeil si PLF était issu du Sénat il n'y aurait par exemple plus de financement des APL ni de financement pour les maisons France service plus de financement pour le logement des des des personnes en difficulté. Nous sommes tous ici d'accord pour maîtriser la dépense publique mais mon groupe ne partage absolument absolument pas les cibles choisies pour les réaliser en votant des économies non structurante. Le déficit s'établirait à 3,7% du PIB. Mais ce chiffre est factice, il reflète tout simplement la suppression sèche de politiques publiques qui sont pourtant essentiels. Cela étant, je tiens quand même à saluer un certain nombre d'amendements adoptés issus de notre groupe qui s'avère positif pour les territoires ultramarins à Wallis et Futuna, qui disposera de 450 millions d'euros supplémentaires pour le remplacement des huit générateurs d'hémodialyse à Mayotte avec la prolongation de la majoration à des seuils de revenus fiscaux de référence en dessous desquels les contribuables modestes ou âgées peuvent bénéficier des allégements de taxe foncière.-- En Guadeloupe, avec une augmentation du tarif d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliqué aux centrales géothermiques électrogène essentiel par exemple pour la commune de Bouillante, sans oublier des mesures plus général comme la prolongation de plusieurs dispositifs de défiscalisation jusqu'en 2029 pour les collectivités d'outre-mer l'augmentation de 4 millions d'euros pour les crédits dédiés à la lutte contre l'habitat insalubre ou encore le relèvement de la franchise de taxation à l'octroi de mer et à la TVA pour les des bien, qui font l'objet de petits envois non commerciaux de 205 à 400 euros de nouveau une mesure de soutien au pouvoir d'achat des ménages, compte tenu de l'adoption de ces amendements qui justifieront le vote positif de mes collègues le tamarin vous comprendrez néanmoins qu'une majorité de notre de notre groupe RDPI s'abstiendra sur ce vote sur le vote de ce projet de loi de finances pour 2023. Merci. Mes chers collègues. Le Sénat va maintenant procéder au vote sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Je rappelle que le scrutin public et de droit. Et conformément à l'article 70 de notre règlement le scrutin public aura lieu à la tribune. Ceux qui souhaitent voter pour. Placeront un bulletin bleu. Dans l'urne placée. À cet effet.

Vos bulletins de vote personnel sont. Vous le savez à votre disposition dans une enveloppe placée dans le tiroir du pupitre. Si vous êtes titulaire d'une délégation de vote. Vous y trouverez également une enveloppe Je vais demander à. 2 collègues secrétaire du Sénat. De m'aider à superviser les opérations de vote. En l'occurrence madame Françoise Férat. Et monsieur Joël Guerriau.

Voici le moment de plus grande incertitude de la journée. Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel nominal. La lettre H.

Monsieur le

Il ne va donc pas être procédé. Nouvel appel nominal puisque. Donc plus personne ne demande à voter.-- Le scrutin est clos.-- J'invite madame et messieurs les secrétaires procéder au dépouillement. Il

Merci. Numéro 94 sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote. Nombre de votants, 347. Nombre de suffrages exprimés. 305. Pour l'adoption, 197 contre 108, le Sénat a donc adopté le projet de loi de finances pour 2023 tels qu'ils résultent de de ces travaux. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous venons d'adopter ce projet de loi de finances au terme. Je donne un peu statistiques mais ça montrera votre présence au banc. 160 heures de séance. Soit 10h de plus. Il y a 2 ans. C'est quand même une durée record. Ce sera pour nos méditations futur. Mes chers collègues en conférence des présidents. Soit une durée record depuis 1995. Avec pardonnez-moi la statistique un nombre record d'amendements. 3057. Je souhaite vraiment remercier le rapporteur général de la commission des finances Jean-François Husson, qui par son travail. En rigueur et en vigueur à éclairer nos débats ces dernières semaines sur l'ensemble des politiques publiques examiner. S'est également félicité le président de la commission des finances Claude Raynal qui, en bon Capitaine a eu parfois et même souvent à choquer un peu nos voiles lorsque l'hémicycle était tenté de le fait un peu. Cela nous a permis malgré quelques coups de vent de naviguer dans une sérénité. J'allais dire de bon aloi pour tenir le calendrier de la discussion budgétaire telle qu'il est fixé par notre Constitution. Je veux saluer tous les autres membres de l'équipage. Je pense bien sûr aux aux 47 rapporteurs spéciaux de la commission des finances au 77, rapporteur pour avis des autres commissions ainsi qu'à leur président au chef de file des 8 groupes politiques au vice-, président et vice-présidente qui ont conduit nos débats tout au long de ces semaines je voulais les remercier. Particulièrement les vice-, président et vice-président. Je voudrais remercier également l'ensemble des personnels des services du Sénat des groupes politiques pour leur disponibilité et leur engagement et permettez-moi de saluer particulièrement. Les collaborateurs de commission qui ont été extrêmement peu raison. Les personnels du Sénat. Qui ont fait face. Je voudrais, Monsieur le Ministre vous remercier. De donner le nombre d'heures pour votre présence assidue. Au cours de l'examen de ce projet de loi de finances pour les conciliabules nécessaires à l'extérieur. De l'hémicycle aussi qui font partie intégrante de la vie parlementaire. Je voudrais avant de donner la parole au ministre, monsieur le président de la commission sur le rapporteur général si vous souhaitiez dire quelques mots. Monsieur le président.-- Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mots après vous. Tout d'abord pour. Pour vous dire 2 choses, la première c'est que j'ai toujours plaisir à ce que l'on termine cette partie se sur le PLF, et le problème de vote sur le projet de haute finance par un scrutin à la tribune. J'y attache beaucoup d'importance. Je sais qu'on y passe peut être une heure que certains pourraient regretter mais je pense que ça donne. À ce moment une force particulière et j'y suis tout particulièrement. Attaché. Vous dire aussi que quand même on y attacher mais certains je dirais Patrice. Je ne dirais pas ça, mais quand même organiser les choses de manière à passer en 1er voyez je ne veux pas citer le rapporteur Husson venant je me permettrai pas, mais c'est la 3ème année d'affilée, que c'est la lettre H que l'on tire un premier. Je voudrais pas voir la malice. Je voudrais pas voilà, mais tout de même c'est quelque chose d'assez particulier, si on fait un petit concours là de regarder combien combien on a de chances que ça soit 3 fois d'affilée. On verra qu'il faut c'est pas mal hein statistique. Bien. Je souhaiterais moi même. Monsieur le Président vous remercier. D'ouvrir de conclure notamment. Nos débats. Ainsi que les vice-président de séance. Comme vous l'avez fait, qui ont présidé à la bonne organisation de nos travaux et je dois dire que cette année. Ce ne fut pas si simple. Ça ne veut pas dire que les années précédentes, c'était très simple mais là c'était quand même très très particulier. Salué évidemment. Notre rapporteur général. Qui est évidemment aux avant-postes durant toute la période. Ainsi que tous les rapporteurs faut spéciaux, rapporteur pour avis l'ensemble des services du Sénat et notamment je le dis, particulièrement ceux de la séance. Parce qu'il a fallu. Comment dire essayer de modifier travailler pour que les débats se passe au mieux et nous aurons sans doute à progresser toujours collectivement sur ce poste. Et puis comme vous saluer. Notre ministre au banc. Gabriel Attal et l'ensemble de son cabinet et de sa disponibilité de son envie également de parler, c'est-à-dire de s'exprimer. D'expliquer ses positions et c'est utile évidemment d'un autre, d'un Vous l'avez dit, monsieur le président. 3000 amendements. Alors je voudrais rerapellé je crois que notre ami Jérôme Bascher la fait tout à l'heure mais quand même hein il y a 10 ans on était à 500 amendements. 500. Il y a 5 ans on était à 1000. On est aujourd'hui à 3000. Oserais-je dire, n'en jetez plus la coupe est pleine. C'est-à-dire qu'après, évidemment notre difficulté c'est de rentrer tout ça dans un temps qui est fixée par la Constitution. Étiez fixé comme vous le savez, à une vingtaine de journée donc ceci s'impose à nous et nous obligera, sans doute dans les mois qui viennent à réfléchir sur effectivement l'organisation de ces travaux pour qu'il se passe au mieux dans le délai contraint par la Constitution. Et c'était inutile de faire tout ce travail, c'est-à-dire 3 mois de travail en commission trois semaines en session. Si évidemment l'Assemblée nationale, le gouvernement avait comme idée de ne pas reprendre pleinement. En compte cette lecture complète au Sénat mais je sais que ils ne vont pas hésiter à le faire et en tire les conséquences en vue de l'adoption du terre du texte définitif dans merci encore un peu de travail mais on va y arriver. Merci. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission. Mes chers collègues, juste quelques mots pour. Moi aussi adressé des remerciements à l'ensemble des sénatrices et des sénateurs et à l'ensemble des équipes du Sénat sur le plateau. Dans les coulisses et puis dans tout le temps qui à la fois précède l'examen du budget, mais également le temps de l'examen du budget ou je le je le confesse volontiers, les nuits sont très courtes. Elle se répète souvent à être très courte mais. Même si c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je dois dire que les uns et les autres. On a trouvé les modalités à la fois de l'écoute de l'échange parfois bref parfois plus développée, je le vous le dis c'est la troisième année. L'an dernier, ça a été plus court cette finalement à la fois c'est une forme de marathon, mais c'est aussi une manière de sentir qu'elle est le le pouls de la France à travers les expressions des uns et des autres dans ma fonction, je m'efforce toujours de. Garder un ton à la fois juste de temps en temps. De mettre une petite plaisanterie parce que même si il faut être sérieux. Il n'empêche que on peut de temps à autre. Trouver des moments de respiration et puis Monsieur le Ministre, je crois que le plus important nous attend. C'est. Ce qu'il reste en sortant ici du Sénat puisqu'il n'a échappé à personne que nous sommes dans un quinquennat d'un temps nouveau, avec une assemblée nationale. Plus complexe en terme de majorité et de gestion et une chambre haute, qui vous donne des messages clairs. Avec des positions assez unanime sur un certain nombre de sujets c'est ni le moment, ni l'heure de vous. Rappeler. Ce qu'on vous propose de porter et de garder dans le débat démocratique, parce que nous devons me semble-t-il, à cette heure prendre garde au moins d'une chose, c'est faire en sorte que le Parlement continue d'être écouté, entendu à la fois par la voix qu'il porte mais par les décisions qu'il prend et qu'il confie au gouvernement, notre responsabilité collective être importante importante parce que on s'apprête à à mon avis à connaître des temps plus difficiles et nous devons être aux côtés des Français pour les aider à traverser. Sans crainte particulière sans. Amplifier les angoisses mais en se donnant la main avec les élus locaux avec les chefs d'entreprise pour faire en sorte que demain en 2023 et dans les années suivantes il fasse encore bon vivre dans notre si beau pays de France. Merci.

Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénatrices et sénateurs à mon tour je veux remercier le président de la commission des finances le rapporteur. Général du budget ses nombreuses heures d'examen et la qualité du travail que nous avons eue ensemble remercier aussi l'ensemble des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis qui ont participé organisée. Contribuer à ce travail qui nous a. Accompagnés pendant plusieurs semaines. Jérôme Bascher disait que c'était le 1er PLF sous l'empire de la nouvelle Lolfe pour moi, c'était tout simplement le 1er PLF en tant que ministre du Budget et donc le premier examen au Sénat et. Je dois dire que j'ai énormément apprécié les échanges que nous avons eu, ils ont toujours été empreint. D'une très grande courtoisie républicaine d'un très grand respect d'une très grande écoute mutuelle et je dois le dire, ça fait du bien ça fait du bien. On a eu de vrais débats. Parfois de vraies divergences dont je n'irai pas jusque là mais en tout cas, en tout cas ça fait ça fait du bien et je pense que c'est utile. Je pense profondément que c'est utile vous adopter aujourd'hui un texte qui est assez sensiblement différent du projet de loi qui vous avez été. Présenté il y a un solde qui s'améliore mais comme l'a dit Emmanuel Capus en trompe-l'oeil puisque c'est essentiellement le fait de ministères et de pans entiers de l'action publique qui sont supprimés. Je pense au ministère de la cohésion des territoires au ministère de l'agriculture à l'action territorial de l'État. Mais ce que je veux dire c'est que si la navette parlementaire nous permettra évidemment de rétablir un certain nombre de suppressions qui ont eu lieu, je crois profondément qu'il restera la marque du Sénat dans le texte qui sera adopté à l'issue de la navette parlementaire. Parce qu'il y a des amendements très concrets, très important pour la vie quotidienne des Français pour monter nos territoires qui ont été adoptés il y en a beaucoup, je peux pas tous les citer mais je pense à l'amendement qui avait été déposée par une très grande partie des bon je crois même l'intégralité des groupes notamment par monsieur Rickman sur la suppression du malus auto pour les SDIS et pour la protection civile. la à la à l'amendement qui majore la dotation biodiversité porté par Bernard Delcros, je pense à l'amendement sur l'habitat insalubre en outre-mer porté par Georges Patient. Je pense à l'amendement sur la continuité territoriale et sur le prix des billets d'avion, porté par Madame Jacques je pense à l'amendement sur les prêts et les avances pour l'Iran et leur suppression porté par monsieur Cosic c'est aussi un élément très important dans le contexte que nous connaissons. Je pense à de très nombreux amendements qui sont très concrets pour nos valeurs ou pour la vie des Français dans tous les territoires et je pourrais en citer d'autres, il y a ensuite des. Grands sujets qui ont irrigué nos débats, je vois le président de la commission. Je pense aussi à ces amendements qui ont été portées sur le financement des nouvelles LGV très important aussi pour nos territoires et la cohésion des territoires, les lignes à grande vitesse et rapporteur général pour citer tout le monde et ces amendements sur la lutte contre la fraude fiscale issu du très bon rapport sénatorial de la commission des finances sur la lutte contre à la fraude. Il reste, je le disais de grands sujets. La suppression de la CVAE. Vous avez souhaité supprimer et là je le dis d'emblée, je l'ai dit après le vote. Nous proposerons à l'Assemblée nationale de rétablir la suppression de la CVAE. Mais j'ai bien retenu de nos échanges que nous pouvions aller plus loin, être plus clair sur les modalités de compensation pour les collectivités territoriales et croyez bien que nous allons poursuivre le travail en la matière pour être plus convainquant sur le sujet il y a ensuite un nouveau filet de sécurité qui a été adopté ici à l'initiative du rapporteur général et de différents groupes, je ne sais pas si le filet qui sera adopté à la fin du processus parlementaire sera exactement celui du Sénat ce que je sais c'est qu'il sera différent de celui qui avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale pour concerner davantage de communes et j'ai bien entendu là aussi le message que vous avez porté pour que davantage de communes puissent être concernés et être accompagné et donc nous tiendrons compte évidemment de ce que vous avez porté y compris dans ce cadre là ici au Sénat, tous les sujets que je viens d'évoquer monte que nous avons abordé des enjeux très concrets pour la vie des Français et de nos collectivités rapporteur général là dit. Notre pays et le monde entier connaît des troubles, des inquiétudes des angoisses. Et je crois que s'il est un élément profondément rassurant dans ce contexte, c'est la capacité à continuer à se parler à travailler ensemble, à échanger des arguments chacun avec nos sensibilités chacun avec nos tempéraments mais toujours dans l'intérêt des Français, c'est ce que j'ai vécu ici ces dernières semaines avec vous, merci à tous. Merci monsieur. Je vais suspendre la séance quelques instants pour permettre à chacun. De respirer un peu, de s'installer pour l'examen du prochain point de l'ordre du jour. La séance est suspendue. Elle sera reprise dans 10 minutes.

La séance est reprise. Alors la parole est à monsieur Claude Kern pour une mise au point, au sujet d'un vote. souhaite modifier son vote du scrutin numéro 51 sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale du 15 novembre 2022. Elle souhaite modifier son vote en abstention au lieu de ne prend pas part au vote, elle vous remercie. Merci acté donner de votre mise au point et elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote en 2ème lecture sur la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale visant à limiter l'an grillage ment des espaces naturels et à propos, à protéger, pardon la propriété privée. Et la parole est à Madame. Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Moi je m'amène la ministre. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le rapporteur. Monsieur le sénateur Jean-Noël Cardoux mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Aujourd'hui est une étape importante pour la biodiversité française. Aujourd'hui vous avez l'opportunité de mettre fin à des années de dégradation de notre belle nature. Aujourd'hui, il vous est offert la possibilité de voter la proposition de loi visant à limiter l'an grièvement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Le gouvernement fait déjà beaucoup pour la biodiversité. Un fonds Vert de 2 milliards d'euros va être déployé 150 millions d'euros seront consacrés à notre stratégie nationale pour la biodiversité. C'est inédit.-- Nous nous étions fixé un objectif de protection de 30% de notre territoire terrestre et marin que nous avons atteint. 10% du territoire sera même bientôt en protection forte nous défendons les mêmes objectifs au niveau international. Nous mettons en place des plans d'action nationaux pour protéger les espèces en danger également. Et je pourrais encore en dire beaucoup sur notre action, cette liste est longue car nous agissons avec détermination. La protection de notre biodiversité passe aussi par l'arrêt et le retrait de ces grillages ils ruinent nos paysages naturels. Il faut que les citoyens qui nous regardent et nous écoutent se rendent compte. En 2019, plus de 3000 kilomètres de grillage au minimum avaient été recensés sur les 3 départements du Loiret du Cher et du Loir-et-Cher. Comment ne pas s'indigner d'un tel chiffre. Cette proposition de loi, c'est la concrétisation d'un bel exemple de coconstruction législative avec le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement que la politique est belle quand elle nous réunit ainsi pour l'intérêt commun du plus grand nombre. Je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'examen de la proposition de loi a commencé ici au Sénat. Monsieur le sénateur Jean-Noël Cardoux vous en êtes à l'initiative et je veux saluer une fois de. Suisse. Votre engagement sincère.-- Sur ce sujet important pour votre belle Sologne. J'en profite également pour saluer le travail des rapporteurs des deux chambres Laurent Somon et Richard Ramos à l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle étape dans l'examen de ce texte après l'avoir examiné la semaine dernière en Lake. Cet examen a été l'occasion d'un dialogue apaisé et constructif le choix du format en Lake témoigne de l'efficacité des débats que nous avons eu. Ce texte atteint de nombreux objectifs que nous partageons. Il met fin à l'grièvement qui rompt les continuités écologiques pour leur suivi les essais, les espèces doivent se déplacer sans contrainte avec la trame verte et bleue. Nous devons reconstituer un réseau d'échange pour que les espèces animales et végétales puissent circuler s'alimenter se reproduire se reposer et ainsi assurer leur cycle de vie.-- Il met fin à la défiguration de notre paysage. Nos concitoyens attendent de nous que nous restions et resterions la beauté de nos campagnes. Nous ne pouvons pas laisser quelques-uns s'accaparer nos bois, nos forêts et nos prairies. Il met également fin à des obstacles qui nous empêche de lutter contre les incendies. Le risque d'incendie grandi dans un contexte de réchauffement climatique. Il touche dorénavant des régions que nous pensions jusqu'à présent épargné. Il est de notre devoir d'aider nos pompiers à accéder facilement à ces zones. Nous sommes évidemment conscient que certains clôtures sont nécessaires, elle protège parfois nos routes et nos voies ferrées. Elle participe aussi à la régénération forestière et soutiennent l'activité agricole.-- Ces clôtures ne seront pas concernées. Celles que nous devons réguler sont celles développées pour des pratiques purement cynégétique ou celles relevant de la propriété privée qui se sont trop largement étendu. De points en particulier dans ce texte mérite d'être souligné. D'abord l'article 1er, il prévoit une obligation de mise en conformité des clôtures hermétique pour rétablir les continuités écologiques lors de la navette parlementaire. Le délai de prescription a évolué le gouvernement il y était favorable. Une prescription de 30 ans a été introduit de manière à ce que la date ne soit pas contestable. Ce point a été sécurisé. Donc, juridiquement il a fait l'objet d'une étude de constitutionnalité qui en a souligné la pertinence.-- En Lake, un point a été soulevé pour s'assurer que les troupeaux et l'agro-pastoralisme était bien compris dans les exceptions. J'ai pu confirmer que c'était le cas je me suis engagé à ce qu'une circulaire viennent explicitement précisé cette cette exception pour lever toute ambiguïté. L'article 5 ensuite. Il est le fruit d'une coconstruction entre le Sénat, l'Assemblée et le gouvernement initialement introduit par les députés. Il prévoyait l'interdiction d'agrainage et d'affouragement dans les espaces clos. Le Sénat est venu préciser juridiquement cette disposition pour définir les espaces clos concernés à savoir les espaces étanches, qui ne permettent pas le passage des animaux non domestiques. J'ai été également favorable.-- Elle permet de rétablir la cohérence entre les espaces ouverts et les espaces clos permettant le passage des animaux domestiques pour lesquels il est clairement précisé désormais que la même réglementation s'applique. Cela va donc dans le bon sens. L'efficacité de notre âme à notre travail et va permettre la mise en place rapide de cette nouvelle législation. Le gouvernement souhaite en effet que le texte que vous vous êtes appelés à voter aujourd'hui soit soumis très rapidement à l'Assemblée nationale en 2ème lecture une fois adopté, il sera nécessaire de poursuive le travail sur le terrain. Il nous faut engager une action efficace qui se concrétise le plus rapidement possible. Le dialogue devra donc débuter très prochainement avec les acteurs du terrain. Les propriétaires, comme les élus, les fédérations départementales des chasseurs comme les associations écologiques ils devons nous assurer que cette transition se déroule dans les meilleures conditions. Je suis convaincu que cette proposition de loi sera une contribution réellement significative en faveur de la biodiversité. J'aurai l'occasion de porter personnellement haut et fort au nom du gouvernement, cet enjeu majeur lors de l'événement international de la COP15 à Montréal. Comptez sur moi pour mettre toute mon énergie et aboutir à une COP décisive avec des objets. Clairs, ambitieux et surtout quantifier associée à des moyens de financement adaptés. Nous agissons en France autant qu'à l'international. C'est ainsi que nous sauverons notre biodiversité. Je vous remercie.-- Merci madame la ministre. La parole est à monsieur Laurent Somon, rapporteur de la commission des affaires économiques pour sept minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre. Madame la présidente de la commission. Mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur la proposition de loi présentée par Jean-Noël Cardoux visant à limiter l'an grièvement des espaces naturels et protéger la propriété privée. Elle a été examinée et votée la semaine passée en deuxième lecture par notre commission des affaires économiques dans le cadre de la procédure de législation en commission. En première lecture cette proposition de loi a reçu l'approbation unanime du Sénat et de l'Assemblée nationale. J'espère qu'il en sera de même cet après-midi. Ce rare et remarquable consensus est le fruit d'une patiente construction. En s'attaquant au fléau de l'emprisonnement de la nature. Ce texte a réussi à rassembler, sénateurs et députés chasseurs et non-chasseurs citoyens et associations, engagé de longue date dans ce combat. Il y avait urgence tant leur grièvement pose des problèmes pour la sécurité dans la lutte contre les incendies. La libre-circulation de la faune et l'attractivité de nos territoires ruraux.-- Cette réussite est en 1er lieu le résultat du travail de l'engagement de son auteur, Jean-Noël Cardoux que je tiens à saluer. Ce texte Ce texte très complet et le fruit de sa grande connaissance de la chasse ardent des fesses défenseur de notre Patrimoine naturel et forestiers. Il a su faire des propositions en dehors de tout esprit partisan. Militant pour une chasse durable éthique exigeante. Il a dénoncé l'artificialisation des pratiques de chasse et de sylviculture ainsi que l'enfermement de la nature comme des hommes derrière les grillages. Sa proposition de loi dès sa rédaction initiale adopter une approche globale et des solutions équilibrées. Dont la pertinence a été relevé par les 2 assemblées. Je tiens également à remercier le député Richard Ramos, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale à l'écoute des différentes sensibilités. Il a su rassembler pour aboutir à un approfondissement des dispositions votées par le Sénat. Sa recherche du consensus est à souligner et manifeste la vente volonté d'avancer ensemble vers l'objectif commun de protection de nos espaces naturels. Je voudrais enfin vous remercier Madame la Ministre pour votre disponibilité et votre aide pour permettre à cette initiative parlementaire d'aboutir. Je veux bien sûr y associer les services de votre ministère ainsi que l'OFB dont l'expertise a été précieuse pour enrichir le texte, je me félicite de ce travail partenarial. L'objectif de la commission des affaires économiques a été de consolider la proposition de loi en garantissant l'équilibre du texte entre d'un côté le désengagement de l'autre le respect du droit de propriété mais aussi en garantissant sa bonne application. Ainsi, en première lecture, la commission avait étendu les pouvoirs de contrôle des agents de l'Office français de la biodiversité, afin de faire appliquer le droit de la chasse. Partout où elle se pratique et plus particulièrement dans les enclos qui ici soustrayez. Elles avaient aussi voulu démultiplier les capacités de contrôle en étendant les pouvoirs des agents assermentés des fédérations départementales des chasseurs. La Commission avait en outre veiller à sortir les dispositions de la proposition de loi d'un volet répressif. En instaurant une sanction pour non respect des nouvelles règles applicables aux clôtures dont vous avez rappelé les modalités Madame la Ministre. En 2ème, lecture, nous avons adopté conforme la quasi-totalité des articles amendés par l'Assemblée nationale. Les modifications restantes en ligne avec les orientations définies par le Sénat en première lecture. L'unique amendement adopté par la commission à l'article 5 sur la réglementation de l'affouragement et de l'agrainage poursuit ce travail de mise en cohérence et traduit une vision une vision commune des solutions à adopter. Madame la présidente. Monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues. Pour conclure je formule le voeu que ce texte soit adopté dès début 2023 à l'Assemblée nationale afin de garantir une application rapide et effective de la loi.-- Je suis heureux de voir un texte dépasser les oppositions partisanes par des compromis constructif entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat dans le but de protéger l'intérêt général. Nous pouvons en être fiers. Pour que les milieux naturels reste des havres de paix et de tranquillité libérons les de ces grillages et ton contrôleur artificialisation. Proton je protégeant leur faune et leur flore qui font leur charme et leur bonheur. Et pour satisfaire à l'envie de lyrisme de François Bonhomme. Avec notre illustres prédécesseurs Victor Hugo préférons au fil de fer Le Havre du génie de la nature je cite je ne demande pas autre chose aux forêts que de faire silence autour des entre frais et de ne pas troubler la chanson des Fauvettes je je veux entendre aller et venir les navettes de pense noir tisserand que nous entrevoyons et qui file en tordant l'eau, le vent les rayons ce grand réseau la vie. Immense et sombre toile où 30 en bas de fleurs en en bas la fleur en haut, l'étoile.-- Et de terminer par une note moins célèbres mais plus personnel voilà cette nature partagés que j'observe vu des chemins autorisés chasseur d'images ou de gibier tous s'engagés à la protéger. Respect du gibier et de la propriété privée, il était urgent d'y contribuer à nous de légiférer. Hé bien après ce moment de poésie. Nous allons entendre Madame Cécile Cukierman. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste chers collègues pour cinq minutes. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, je m'en excuserez, je ne vous ferai pas une intervention ni en alexandrins ni rime mais finalement sur un exercice qui peut lui aussi prend tout son sens qui est celui de la prose libre. Bien je pour revenir sur notre texte et comme nous l'avions rappelé lors de la première lecture ici au Sénat, cette proposition de loi qui vise à garantir cela a été dit la libre circulation des animaux sauvages dans le territoire concerné par les pratiques grièvement et pour nous. Bienvenue. Si ce phénomène n'est pas nouveau, il n'est plus circonscrit à la seule Sologne et concerne aujourd'hui de plus en plus de territoire. Le président de la Fédération nationale des chasseurs disait lors d'une assemblée qu'il s'agissait d'un vrai problème, c'est un vrai sujet, parce que si on ne bouge pas rapidement, on va finir par avoir des caches partout en France. En effet, cette pratique qui fait obstacle aux continuités écologiques pose des problèmes de sécurité incendie et de sécurité sanitaire empêche la libre circulation de la faune cantonne les populations de gibier à l'intérieur de domaine interdit la promenade nuit au développement du tourisme rural mais elle 3 d'lui aussi une logique de privatisation de nos espaces forestiers qui en exerce serbe les conflits d'usage. Comme le souligne le rapport de la mission d'information sur le grillage m'en Sologne. Il s'agit d'une appropriation renforcé de l'espace, un frein à l'exercice de la police de l'environnement par une déviance du droit des enclos créant des zones de non-droit où la gestion cynégétique est devenue aberrante. Le rapport mentionne même des installations de miradors de poste de tir mettant en danger les usagers de voie publique. Loin donc d'être un texte contre la chasse. Cette proposition de loi met fin à une pratique. Réservée à une très petite partie de la population à une élite qui pouvait s'apparenter plus à un carnage. Et je veux le dire ici, ce n'est pas là le sens de la chasse. N'en déplaise à certains. De plus, ces barrières entraîne des risques sanitaires. Je l'ai dit surdensité mais émettrice des populations elles interrogent sur l'égalité d'application du droit de la chasse sur l'éthique, ainsi que sur l'illégalité de certaines pratiques, comme le souligne le rapport commandé par le ministère de la transition écologique en 2019. En ce sens la chasse en enclos contrevient au principe même d'une chasse populaire issu de la Révolution française finalement d'un acquis de fait de la République. En étendant le droit commun de la chasse à l'ensemble des territoires sur lesquels celle-ci est pratiquée et en renforçant la. C'est aux enclos cynégétique à des fins de contrôle. Cette proposition de loi marque une avancée significative. Même si nous pouvons regretter que le texte n'aille pas jusqu'à interdire la chasse en enclos à caractère commercial. Toutefois, nous regardons comme une avancée la possibilité des désormais désormais pardon aux fesses offertes aux gardes de l'OFB d'aller voir ce qui se passe dans ces enclos sans avoir à saisir le juge des libertés et de la détention en cas de refus du propriétaire.-- De plus, nous nous réjouissons de l'équilibre trouvé entre les deux chambres. Quant à la sanction en cas de pénétration dans la propriété rurale forestière puisque ne sera sanctionné par une contravention de 4ème classe la violation d'une propriété uniquement dans le cas où le caractère privé du lieu est clairement identifié par une signalétique spécifique le débat et la navette parlementaire ont donc conduit à ce texte qui ne paraît prendre la bonne direction qui nous paraît être aussi un des éléments pour. Et c'est le voeu que nous pouvons faire en cette fin d'année tenter d'apaiser le plus et le mieux possible le débat autour de la chasse dans notre dans notre pays facilité et permettent s'être pratique sans. Accompagner les excès. Je crois que attendu effectivement par les chasseurs et les différents acteurs de nos territoires ruraux. Cette proposition de loi va dans le bon sens et nous la voterons.-- Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Paul Prince pour l'Union, l'Union centriste et pour cinq minutes. Madame la présidente. Madame la ministre. Madame la présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens as tout d'abord à réitérer mes remerciements à notre collègue Jean-Noël Cardoux pour avoir permis à ce sujet clé pour nos territoires d'être inscrit à l'ordre du jour de notre chambre. Ce texte contribuent de continuer à faire du Sénat d'une véritable caisse de résonance des d'enjeux territoriaux. Cette proposition de loi, témoigne également du travail long et minutieux de notre collègue, rapporteur du texte, Laurence homos qui a su s'emparer du sujet lors des 2 lectures afin de faire évoluer le texte pour le rendre encore plus complet juridiquement et lui donner une ampleur qui a su convaincre les membres de la chambre basse de notre Parlement. J'en profite pour saluer leurs travaux et notamment à l'implication du rapporteur Richard Ramos sur ce texte qui ont permis de corriger certaines malfaçons et de mètres cette proposition de loi toujours plus en adéquation avec la rééditer de nos territoires.-- Le grillage moi des espaces naturels est un phénomène déjà ancien, mais qui a tendance à s'accentuer et a contaminé si j'ose dire une part de plus en plus important de notre territoire.-- La Sologne souvent pris en exemple et malheureusement caractéristique de ce phénomène. Comme d'autres ici je la connais bien et même très bien. C'est ainsi qu'aujourd'hui. On y compte près de 4000 kilomètres de grillage. C'est plus que le nombre de kilomètres de routes départementales, dans mon département de Loir-et-Cher. Un chiffre révélateur des dérives néfastes de un grillage moi. Le développement de celui-ci est un des symboles de l'évolution de la ruralité dans notre pays mais aussi de l'accroissement d'une forme d'égoïsme dans notre société. Il caractérise non seulement une défense excessive du droit de propriété et un manque de respect des terrains d'autrui mais aussi une perte de la culture rurale et cynégétique ainsi qu'une atteinte à la biodiversité. Cette proposition de loi visant à limiter leurs grillage moi des espaces naturels et à protéger la propriété privée que nous examinions en seconde lecture souhaite poser des règles pour mettre fin à ces difficultés. Avec pour conséquence l'amélioration de la sécurité incendie, la protection de la sécurité sanitaire, l'arrêt de la destruction de la faune et de la flore, ainsi que le développement du tourisme rural. Le dispositif proposé et globale et les mesures vont dans la bonne direction. L'interdiction des clôtures, qui ne laisse pas passer la faune et qui utilise des matériaux naturels représentent le coeur de ce texte. Il s'agit finalement de redonner de l'air à nos ruralité et à nos forêts sans priver les propriétaires de leurs biens. Le renforcement du volet pénal condamnant les intrusions dans les propriétés privées et salutaire afin de donner des garanties aux propriétaires est équilibré. Le texte. Enfin, l'obligation de mise en conformité des clôtures d'un temps de moins de 30 ans et non plus en 2005 après examen de l'Assemblée. Preuve de l'intérêt pour le Parlement de travailler de concert au service de nos territoires permettra de contourner le phénomène d'opportunités que l'on a pu constater visant à grillager rapidement par peur de la nouvelle réglementation. Les exceptions prévues et recalibrer par les rapporteurs des 2 assemblées sont aussi importantes à l'image de la prise en compte du caractère historique et patrimoniale des clôtures. Cependant, j'attire votre attention, mes chers collègues, sur une nouvelle disposition introduite à l'Assemblée nationale, qui à mon sens est problématique l'interdiction de la pratique de l'agrainage et de la fourrage mondain en enclos. Je ne suis pas favorable à cette interdiction aussi rigide que dogmatique. Ne s'inspire pas de la réalité du terrain mais les récents rapports de la commission des affaires économiques élaboré grâce à la procédure de législation en commission me semble aller dans le bon sens. En conclusion, vous l'aurez compris, bien que j'une réserve sur les dispositions relatives à l'interdiction de l'agrainage et de l'encouragement. Je soutiens pleinement le texte de cette proposition de loi et la majorité du groupe Union centriste votera en sa faveur. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean Louis Masson 3 minutes.

Madame le président, madame le Ministre, chers collègues. Je crois je considère que cette. Ce cette loi que nous sommes en train d'adopter est un texte excellent. Car de toute manière, nous ne pouvions pas continuer à laisser. Là l'ensemble de la France. Se faire ont grillagé et. Privatisé, on ne pouvait pas laisser privatiser tous les espaces naturels.-- On a assisté. Ces dernières années à une explosion de cet accaparement de l'espace public des forêts et je crois que c'est une très très mauvaise chose. Il y a eu une navette entre l'Assemblée et le, l'Assemblée nationale et le Sénat et cette navette à apporter des améliorations substantielles. Ce dont je me félicite, c'est que. Finalement. Nous avons maintenu quand même les enclos qui existait depuis très longtemps et c'est je pense que les ces enclos qui existait depuis très longtemps, qui ont pour certains une dimension historique. Était en fait victime au niveau du discrédit de ce qui se fait depuis une dizaine d'années de manière tout à fait abusive et contre quoi il fallait réagir, donc. Ce travail en commun entre l'Assemblée nationale et le Sénat a été très porteur puisque nous avons sont bien. Ce qui se passe en Sologne. Parce que le plus mauvais exemple enfance mon la Sologne mais c'est vrai quand on voit les chiffres c'est quelque chose de tout à fait effarant ce qui se passe en Sologne et tout à fait scandaleux et il était absolument nécessaire de réagir

est existant depuis un certain nombre d'années. Pourront être maintenus et c'est d'autant plus admissible cette dérogation que finalement ces enclos, ne sont pas si nombreux que cela. C'est seulement dans la période récente, qui a eu cette explosion et contre laquelle il faut réagir. Donc pour ma part, je voterai pour ce projet de loi pour cette proposition de loi.-- Merci beaucoup. La parole est à monsieur Christian Bauby. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes, chers collègues.

Madame la présidente. Madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. La proposition de loi visant à limiter l'un grillage m'des espaces naturels et à protéger leur propriété privée reviennent devant notre Haute assemblée deuxième lecture. suis et par les députés dans le fin de fonds d'élargissement. Son objectif est de stopper l'expansion de leur pratique de la grille largement. Aujourd'hui 3 ou 4000 kilomètre linéaire de clôture. Érigée sur des propriétés privées. Empêchant à la fois la circulation de la faune sauvage sommes brassage génétique. Et une gestion équilibrée de la biodiversité diversité de nos territoires.-- La chasse, donne une image de la chasse. Loin d'être étiqueté. Avec des animaux engraissés tué ça limite le nombre toute l'année sur des propriétés privées. Ce n'est pas Marco absurde de la chasse. Il était urgent de mettre fin aux privilèges de l'enclos. L'article L 424 3 du code de l'environnement distingue de situations de chance sur les propriétés privées. Première Malincourt cynégétique. Apparenté au domicile avec droit de chasse dérogatoire.

Deuxièmement, les établissements de professionnels de chasse à caractère commercial au de chasse. Sauvetage tentant de supprimer ce privilège et encadrer les clôtures érigées dans les. Parcs de chasse dans son article 1er modifia la trame verte. L'Arctique L 371 1 du code de l'environnement et modifié pour réglementer les clôtures qui devront désormais remplir plusieurs conditions. Permettra de tout temps, La Libre cher Kula des animaux sauvages. Ne pas être enterré dans le sol ou dépasser un mètre 20 de hauteur. Être constituées de matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le train, Je suis satisfait que l'Assemblée nationale le qui élargit le périmètre d'application de nos seules de nouvelles règles. Aux zones naturelles et forestières identifiés par les plans locaux d'urbanisme. Ou à défaut. Dans les espaces naturels des trames vertes ne couvre pas tous les espaces protégés subissant un grillage.-- Les clôtures désormais autorisées sont celles qui sont posées autour de parcelles agricoles pour préserver les récoltes ou nécessaires à la protection des régénération forestière. Ainsi que les clôtures d'intérêt public. Concernant la mise en application pour les clôtures résistante au 1er janvier 2021. L'Assemblée nationale a avancé la date limite de mise en conformité au 1er janvier 2027. Ce qui va dans le bon sens, ajoutant 2 ex-champions les clôtures érigées dans un cadre scientifique les domaines nationaux aux chaleur réalisée avant la publication de la loi de 2005 sur le développement des territoires ruraux. La preuve, de 24. Par tous les moyens. Au hein c'est l'extension aux clôture ont réalisé moins de 30 ans avant la publication de la loi de l'obligation de mise en conformité avec les normes environnementales de protection des paysages. Les députés ont estimé que la date de 2005. Limiter les effets de la loi. La majorité des clôtures éthique ayant été édifié dans les années 80. L'article 1er qui prévoit des sanctions pénales en grillagé ou ne pas mettre en conformité la clôture sera puni de 3 ans de prison et 150.000 euros d'amende. L'article 1er sexy prévoit le contrôle par les agents des fédérations de chasse de la conformité des clôtures et des plans de gestion des enclos.

Après de longs débats à l'article 5, ils ont interdit la grenaille l'encouragement jardin clos et dans les espaces naturels défini sur à visée scientifique. Interdiction assoupli par un amendement du rapporteur en commission au Sénat prévoit alerter du choc de ces pratiques dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques sauf exception inscrite au schéma départemental de gestion cynégétique renvoyant au décret d'application. Avec mon groupe, je voterai en faveur de ce texte comportant des avancées répondent un grade de partie aux attentes que j'avais exprimée, ici même, lors de l'examen du texte en première lecture. Merci cher collègue.

Madame la présidente, madame la ministre. Madame la présidente de commission. Monsieur le rapporteur. Chers Laurent poète, poète à ses heures. Nous sommes à la fin du chemin. Presque. Et encore une petite étape à franchir. Nous sommes à la fin du chemin. Et je voudrais même si c'est des redites. Résumé les 3 grands axes qui ont guidé notre réflexion ma réflexion sur ce texte respect des équilibres naturels et de la biodiversité en permettant la libre circulation de la faune sauvage. 2ème. Le respect du droit de propriété. Et 3ème Max qui est tout aussi important. Retour vers une chasse naturelle dans laquelle l'éthique l'emporte sur la performance. On assimile toujours chassé tire c'est une grande erreur. C'est pas parce qu'on tire bien qu'on chasse bien. Mais ça a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de d'incrédulité. Vous n'y arriverez jamais il y a encore peu de temps, on me l'a dit, vous n'y arriverez pas, puis des oppositions. C'est pas par hasard qu'en même temps. On m'a traité d'un côté de bolcheviks et de l'autre de défenseurs du grand capital. Donc je crois que c'est un équilibre et que c'est la traduction que ce texte est équilibré on en parlait depuis longtemps et le Sénat. À son habitude, puisque le Sénat a la réputation d'être une chambre de réflexion qui prend son temps, qui prend du recul. Eh bien tout le monde en parlait. Tout le monde gesticulait tout le monde affichait tout le monde communiqué depuis quelques années. Nous, on a réfléchi, on a étudié et on a. Travaillé plutôt que déclarer et d'afficher. Alors nous touchons maintenant au but grâce à un étroit, travail en commun avec l'Assemblée nationale et le gouvernement. Madame la Ministre. Nous nous sommes découverts puisque vous êtes arrivé il y avait eu d'excellents contacts avec. Madame bah. Et vous avez pris au pied levé la suite toujours dans ce même esprit constructif et je tenais à vous en remercier. Il faut souligner aussi que c'est pas si fréquent de voir des textes, des propositions de loi. Qui ont fait. A été approuvé à l'unanimité aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. C'est pas si fréquent pour les compter. Nous avons à nouveau obtenu l'unanimité en lecture en commission la semaine dernière. Alors chers collègues. Une 4ème unanimité aujourd'hui ça serait parfait pour montrer le chemin de la dernière lecture à l'Assemblée sur l'article 5. Puisque tous les articles ont été con voté conforme. Il faut dire que les améliorations dont certains orateurs ont ont ont parlé il y a quelques instants, ont toutes été négocié avec le rapporteur du texte à l'Assemblée. Richard Ramos, ceux que je connais bien, il est de mon département, il m'a proposé d'inscrire ce texte dans une de ses niches et bien sûr, j'ai accepté. On a travaillé de manière très étroite et toutes les avancées qui ont été votées à l'Assemblée nationale ont fait l'objet d'une concertation entre Richard Ramos et moi, et je pense que lui et moi pouvons en être satisfait. Alors. L'article 5, on en a parlé, il y avait une discrimination de certains territoires. Il y a le problème aussi. J'en peux le prince a souligné. Des territoires complètement clos mais il y a encore pas mal de travail en aval. Beaucoup de décrets d'application à prendre. Sur l'affouragement et l'agrainage mais sur d'autres textes aussi et ce sera une étape que nous allons commencer en concertation avec vos services madame le Ministre bientôt. Alors espérons que cet article 5 puisse être votée très vite à l'Assemblée nationale. Ces quatre lignes 4 lignes si l'Assemblée nationale adopte aussi la lecture en commission, je pense que ça pourrait être fait très vite car tout le monde l'attend. Alors maintenant ben bien sûr. Dans son remerciement. Je vous remercie. Le gouvernement je réitère mes remerciements Madame le Ministre Richard Ramos. Dont on a beaucoup travaillé ensemble. Laurence. Notre rapporteur poète. Qui n'est pas chasseur, mais qui est originaire d'un pays d'un département. Où la chasse est est une institution. Mathieu Meissonnier et l'administrateur qui nous a beaucoup aidé. Qui le permanent si je ne sais pas si on peut s'exprimer comme ça. Du groupe chasse donc il nous a beaucoup intervenue Annie Charlet ce qui doit être dans les tribunes qui est l'ancienne. Responsable juridique du service de l'ONCF. Qu'il a apporté une contribution fondamentale à la rue d'action de ces articles et puis aussi mes collaborateurs et ils sont dans les tribunes, ils se sentent visés. Ça a été un travail d'équipe de doit conclure en disant que, de ce travail. Intense, hé bien il y a pas de vainqueur, c'est simplement la biodiversité et la faune sauvage qui en sortent vainqueurs. Merci beaucoup, cher collègue. La parole est à monsieur Franck Menonville pour le groupe les indépendants pour cinq minutes.

Ce travail intense et ce travail consensuel. Ce texte très attendu et largement soutenue par les associations et notamment la Fédération nationale des chasseurs. Il s'agit là d'un texte important et courageux dans la qualité, c'est aussi ressenti lors des échanges en commission ce travail constructif collégiale et transpartisan et couronnée de succès avec l'adoption à l'unanimité de ce texte en première lecture dans nos 2 assemblées. Je tiens également à souligner le travail de notre rapporteure. Laurenceau. Ensemble, nous nous sommes accordés sur des mesures justes équilibrés pour réguler et limiter le développement de l'an grièvement. Pratiques néfastes et pourtant en pleine expansion est particulièrement répandu en Sologne mais pas que. Et au plus de entre 3000 et 4000 kilomètres de clôtures. Ont été érigés. Une région dont la beauté a été décrite par le prix de Goncourt donc Maurice Genevoix et dans la voix résonne encore dans mon département de la Meuse pour d'autres raisons. Dans son ouvrage, Lio qui dépeint la Sologne ses étant ses chaume et la fulgurance des odeurs.

Plusieurs modifications notables ont été introduites par l'Assemblée nationale, je pense notamment à la rétroactivité qui a été fixé à l'année 92 concernant donc la mise en conformité des clôtures. Il est fixé une date butoir, donc du 1er. Janvier 2027, lui assurant donc une solidité. Juridique. L'Assemblée nationale a également remanié le texte en y ajoutant donc un article 5 qui interdit l'agrainage et la fourrage vend des enclos. Cette disposition soulève cependant une difficulté en effet elle. Introduit une iniquité entre les territoires déjà ouvert et ceux qui le sauront avec la nouvelle loi et cela a été corrigé donc en commission par un amendement du rapporteur qui confirme le principe d'interdiction et qui aménagent donc des exceptions. Encadrés par des décrets qui viendront. Ces évolutions me paraissent aller dans le bon sens et. Et témoigner donc. De débat serein et constructif avec son ensemble des profs forces politique et qui font aujourd'hui. Honneur au Parlement. La proposition de loi donc adopté en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale garantit la liberté de circuler tout en mettant l'accent aussi sur la protection de la biodiversité et en protégeant également le droit de propriété. Elle réussit le défi de préserver de présenter donc une proposition équilibrée entre défense de la propriété privée et lutte contre l'en grillage vend des espaces naturels en effet ce texte Sanctuary.

Il est important de rappeler que la forêt et le foncier agricole ne sont dont aucune manière. Des. Des biens communs mais bien détenus pour 100 dans. Par des propriétaires. Et le fait donc de l'engagement. Le produit est le fruit de l'engagement et du travail des hommes. La proposition de loi donc, permet donc aussi de répondre aux problèmes causés par les pratiques abusives de l'engrais cela crée de de graves difficultés, notamment en matière sanitaire, l'absence de brassage entre les espèces. Qui ne peuvent plus circuler engendrent des hausses de con de consanguinité et des maladies et enfin la prolifération des clôtures induit donc des risques en matière de sécurité incendie puisque les pompiers. Se retrouvent parfois dans l'impossibilité d'accéder à certaines parcelles. Le réchauffement climatique que nous vivons nous rappelle donc à ces gens je donc pour toutes ces raisons, notre groupe se prononce bien évidemment en faveur de ce texte et des modifications portées. Par la commission. À l'issue donc de du débat au Sénat et à l'Assemblée. Merci.-- Merci la parole est à Monsieur Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes.--

Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. Nous avons toutes et tous. Unanimement fait le constat que l'embrayage est un véritable fléau pour nos territoires ruraux et pour la faune, tant il entra il entrave la libre circulation des animaux et entraîne souvent une surpopulation artificiel de gibier. Laquelle provoque des problèmes sanitaires et des effets négatifs pour tout l'écosystème aussi bien la faune que la flore.-- Je me félicite donc aujourd'hui de cette proposition de loi et du travail constructif d'amélioration menée de concert par l'auteur du texte et les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale.-- J'avais proposé en première lecture un amendement malheureusement rejeté visant à réduire le délai de mise en conformité de 7 à 5 ans finalement un délai de 4 années, a été retenu. C'est une excellente décision qui permettra ainsi une application rapide du présent texte, démontrant ainsi une véritable volonté d'agir. Il restera toutefois les enclos antérieurs à 1992. Ce que nous ne pouvons que regretter.-- À part bien entendu les les enclos on va dire patrimoniaux. Je me félicite également d'introduction dans le texte de la traduction d'interdiction de l'agrainage et de la fourrage ment dans les enclos hermétique une interdiction plus générale aurait été préférable même si je comprends que cette technique puisse perdurer exceptionnellement dans une logique de protection des cultures. J'attire toutefois votre attention. Madame la ministre sur les exceptions. Qui seront encadrés par décret qui devront être strictement limitée. N'oublions pas que le nourrissage participe de l'explosion démographique des populations de grands gibiers qui prolifèrent et qui. Ensuite leur chasse car devenus de véritables nuisible. Enfin se pose la question des contrôles, comment s'assurer que l'agrainage l'affouragement ne seront plus pratiqué dans ces enclos. Qu'il s'en assurera. C'est une véritable question. J'en viens aux quelques bémols que contiennent ce texte tout d'abord l'article 2 qui porte la création d'une contravention de 4ème classe pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière. Si l'ajout d'un critère de matérialisation physique des limites d'une propriété privée permet de prévenir tout risque d'infraction involontaire. J'ai été alerté sur le fait que les chasseurs pourraient continuer à pénétrer sur des propriétés privées, au prétexte du passage des chiens de chasse ainsi que leur récupération. Il faut éviter à tout prix qu'on ait un 2 poids 2 mesures c'est dessus situation pourrait générer des conflits aussi un éclaircissement sur ce point semblerait nécessaire. Enfin ce texte de fait l'impasse sur la chasse commerciale on a on enclos de manière générale. Je pense que nous ne pourrons pas esquiver ce débat quant à cette pratique jusqu'alors méconnu mais qui n'est pas pour autant anecdotique, elle concerne, je le rappelle, environ 1300 parc et en cloud qui détiennent au total. 50.000 à 100.000 animaux. Il s'agit en majorité de cerfs de chevreuils, de mouflons et dedans. C'est la question de l'éthique de cette pratique qu'il faut se poser. Je sais que l'auteur de cette proposition de loi est très attaché à l'éthique de la chasse et je pense que là il y a un vrai sujet. 500 euros pour tirer sur un mouflon ou 600 euros pour abattre hein Le sanglier lui côté autour de 300 euros. C'est Safari organisé sans aucune logique de régulation ne sont plus acceptables. Aujourd'hui, il faudra nous y pencher.-- Malgré ces quelques réserves. Le texte porte des évolutions indéniable et je remercie une nouvelle fois son auteur. Il participe à la fois d'une reconquête du paysage et de la libre-circulation de la faune sauvage. Le groupe écologiste soutiendra. Lorsque des jours sans chasse auront été dicté nationalement le retour à la sérénité aura fait un grand pas dans nos forêts et son dress chemins ruraux. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Patricia Schillinger pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour cinq minutes.-- Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, dès le début de l'examen de ce texte au mois de janvier, nous avions été nombreux sur ces bancs, a souligné la menace potentielle de que constitue la pratique de l'an grillage ment pour la bio diversité et plus largement les problèmes environnementaux qu'elle suscite en limitant voire en empêchant la libre circulation de la faune sauvage l'grillage ment entrave la satisfaction par les différentes espèces de leurs besoins écologiques essentiel. Cela peut nuire à leur reproduction ou à l'inverse à l'intérieur des parcs et on et en cloud conduire à une sur-concentration d'espèces favorisant l'accroissement des risques sanitaires ou encore menacé la flore depuis la dernière fois que nous ne sommes penchés sur ce texte. La France a connu une importante vague de chaleur directement imputables au réchauffement climatique, elle s'est traduite dans plusieurs régions par des incendies de forêt, d'une ampleur inédite. Si la problématique de l'an grillage en est intimement liée à la pratique de la chasse. Ces récents événements légitimement d'autant plus la nécessité d'encadrer ce phénomène tend la présence des clôtures peut s'avérer être un frère, un frein à l'intervention des services de secours avec mon groupe RDPI nous tenons à saluer l'esprit de coconstruction dans lequel a été menée l'examen de ce texte pour arriver à une proposition qui parvient à concilier les différents intérêts qui sur ce sujet pouvaient sembler un conciliable. Le gouvernement en coordination avec l'auteur de cette proposition, monsieur le sénateur Jean-Noël Cardoux et notre rapporteur Laurent Somon pour le Sénat ainsi que François Cormier Bouligeon et Richard. Ramos pour l'Assemblée nationale ont su faire évoluer efficacement ce texte de points, on fait plus particulièrement l'objet de discussions, la question de la diff, définition des clôtures qui seraient visés par l'obligation de mise en conformité et celle de l'agrainage et la fourrage ment en sur la première question. Les deux chambres sont parvenus à un consensus autour de la date de 1992. Cette date n'entraîne pas de remise en cause fondamentale du droit de propriété puisque les propriétaires non concernés par l'obligation de mise de conformité son support. Bénéficier de la protection de la prescription trentenaire sur la question de l'interdiction de l'agrainage en espace clos. Celle-ci a été légèrement modifié par notre rapporteur confirmant et précisant le Champ d'application de l'interdiction en envisageant la possibilité d'exception qui seront dessinés par décret. Hormis cette précision, le Sénat a approuvé. Les avancées qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale, ce qui nous laisse espérer une entrée en vigueur rapide du texte pour que ces espaces forestiers trop longtemps défiguré puisse enfin entamer un nouveau chapitre avec les sénateurs ethnies RDPI nous voterons donc pour ce texte, porteur d'une avancée significative en faveur de la biodiversité. Ça Lyon, encore une fois le travail réalisé par son auteur, ainsi que par son rapporteur, tous ont avancé de façon de façon pragmatique, animé par un seul objectif, redonner du sens à la forêt afin, entre autres, de préserver des joies aussi simple que celle de pouvoir librement traverser sans entrave, ces espaces sauvages, merci. Merci la parole est à monsieur Christian Redon s'Arazi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes.

Chers collègues, nous avons été amenés à examiner en seconde lecture selon la procédure de législation en commission la proposition de loi visant à limiter l'grièvement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, preuve qu'elle répondait à une problématique. Sur de nombreux territoires. Elle est devenue un texte transpartisan soutenue par plusieurs groupes politiques du Sénat où elle a été adoptée à l'unanimité en commission et en séance publique, en première lecture. Elle a connu le même sort à l'Assemblée nationale. Nos collègues députés ont néanmoins apporté quelques modifications qui si elles ne remettent pas en cause l'état l'esprit du texte voté au Sénat ont nécessité un nouvel examen de ce texte. Pour rappel, cette proposition de loi émerger en réponse au développement incontrôlé des clôtures en milieu naturel. Autrement dit-il en grillages. Singulièrement sur le territoire du pays de Grande Sologne qui rompt avec l'obligation pour les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels d'assurer la libre-circulation de la faune sauvage, dans le cadre des trames vertes et bleues. De plus en plus de propriétaires installent des enclos de chasse sur leurs parcelles via l'édification de clôture de plus d'un mètre 80. Imperméable au passage de l'homme et des animaux, outre qu'ils. Dégradent le couvert forestier ces enclos nuisent à la continuité écologique et à la biodiversité ne respectant pas les usages locaux comme le spécifier. Le rapport d'août 2019 du conseil général de l'environnement et du développement durable et du conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux ces enclos hermétique je cite sont un non-sens cynégétique et échappent partiellement au contrôle des élus de l'et de l'État sur des interprétations juridiques discutable. Il s'agit bien là de pratiques d'accaparement de privatisation et de perturbations de l'espace naturel et publique qui heurte aussi bien les usagers et les élus que les chasseurs eux-mêmes ces espaces permettant la pratique de la chasse sans interruption saisonnières sans contrôle possible des agents de l'OSB de l'AFB sans plan de chasse sont donc des zones de non-droit qui privatise des espaces issus de notre Patrimoine commun la prolifération de ces parcs de chasse privée était devenue intolérable et démontrer, bien que les seules dispositions du code de l'urbanisme via les PLU ou les paie lui était insuffisante pour permettre aux maires ruraux de lutter contre leur édification. Il nous fallait donc légiférer pour les doter de l'arsenal législatif nécessaire en seconde lecture, l'Assemblée nationale a ainsi précisé un certain nombre de dispositions sans revenir fondamentalement sur sa philosophie. L'article le 1er a été sensiblement enrichie. Outre la précision apportée sur le type de clôture interdite autorisé son Champ d'application est désormais élargie à toutes les zones naturelles et forestières et non seulement celles situées dans une trame verte et bleue.-- le délai de mise en conformité passera donc de 7. Ans avancées obtenues par le Sénat contre 10 ans qui était prévu dans le texte initial la PPL à cinq ans désormais autre avancée ces nouvelles règles s'appliqueront clôture édifié dans les 30 années précédant la promulgation de la présente loi cette extension de prescription permettra ainsi de mettre en conformité, un plus grand nombre de parcs de chasse. En revanche il reste permis de s'interroger comme je l'avais déjà évoquée en première lecture sur qui appréciera l'antériorité de la clôture, l'administration, le maire de la ou des communes concernées. Les risques de connivence avec le propriétaire sont une possibilité qu'on ne peut exclure. Il y a là un flou juridique sur lequel le Parlement n'a pas su répondre de points restent encore sujet à réflexion donc l'Assemblée nationale a introduit un article 5 qui a déjà été largement évoqué et qui vise à interdire l'agrainage et la forage en enclos il modifie le code de l'environnement, en précisant que l'agrainage l'affouragement sont interdits dans tous les espaces clos cet article prévoyait initialement 4 exception la recherche scientifique, la protection de cultures le maintien du bétail. L'établissement de chasse possédant un enclos en séance publique. Seule l'exception pour l'agrainage et l'affouragement menée dans un quatre scientifique a été finalement retenue par les députés dans sa rédaction actuelle cette interdiction aura donc une portée assez large que le rapporteur a néanmoins souhaité redéfinir. J'émettrai quelques réserves sur d'autres points, en particulier les dérogations prévues à l'article 1er, l'Assemblée nationale a maintenu les dérogations porte. Au nombre de neuf qui les porte le nombre de neuf, j'en citerai 2 parmi ces neufs les clôtures des parcs d'entraînement de concours ou des preuves de chaînes chasse et celle nécessaire au déclenchement et à la protection des régénération forestière pour ces exceptions. Comment s'assurer qu'une part certes déclarer comme parc d'entraînement de chasse ne peut de de chasse ne peut pas être détourné de son usage originel et transformé en parc de chasse. Combien de temps mais j'entends une clôture liée à la régénération forestière qui s'assurera. De sa conformité avec la présente quoi comme toujours c'est la question du contrôle et des moyens afférents qui se posent donc hormis ces quelques réserves mon groupe politique souscrit à la position du rapporteur qui propose un vote conforme sur l'ensemble des articles à l'exception de l'article 5 qui demeurera donc le seul restant dans cette navette parlementaire. Il reste beaucoup de questions en suspens sur la mise en application de la présente loi. loi. Félicitons-nous d'avoir déjà pu dans les gares de grandes avancées pour encadrer cette dérive d'accaparement de l'espace public et naturelle et en conséquence, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de ce test. Merci beaucoup. La proposition de loi visant à limiter l'an grillage ment des espaces naturels et à protéger la propriété privée qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. La proposition de loi est adopté. adopté. Je vais suspendre la séance, quelques instants. Pour permettre à chacun de s'installer pour l'examen du prochain point à l'ordre du jour, pense que la séance est suspendue pour cinq minutes.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi sur le déroulement des élections sénatoriales. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Et la parole est à monsieur Stéphane Le Rudulier, rapporteur de la commission des lois pour 7 minutes. la la la présidente madame la Ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par le président François Noël Buffet vise un objectif clair il s'agit de remédier aux difficultés constatées. Lors du scrutin sénatorial de septembre 2020 et ainsi de garantir à l'avenir le bon déroulement des élections sénatoriales. Comme vous le savez, la loi de 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral a étendu aux élections des sénateurs, l'ensemble des règles applicables en matière de propagande électorale aux autres scrutins. Cette loi est entrée en vigueur en juin 2020, si bien que les élections du 27 septembre 2020, ont été le 1er scrutin concerné par son application. Or ce scrutin a révélé de types de difficultés. Des interdictions relatives à la communication des résultats d'une part et à la propagande électorale. D'autre part. En effet, je rappelle que l'article L-49 du code électoral interdit de mener toute action de propagande. La veille, ainsi que le jour du scrutin, tandis que l'article L 52 tiré de interdit de communiquer les résultats de l'élection en métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. L'application de ces 2 articles s'est révélé problématique dans le cas des élections sénatoriales qui sont les seules élections et c'est leur singularité où peuvent avoir lieu de tours de scrutin dans la même journée dans les circonscriptions où l'élection se déroule se déroule au scrutin majoritaire qui correspondent aux circonscriptions dans lesquelles sont élus un ou deux sénateurs c'est-à-dire 52 circonscriptions à l'échelle nationale, le 1er tour de scrutin est ainsi ouvert. De 8h 30 à 11h, tandis que le second tour est ouvert, le cas échéant, de 15h 30 à 17h 30. Dans ces départements, les candidats qualifiés pour le second tour se sont donc trouvés dans une situation pour le moins incongru puisqu'il aurait été strictement interdit de faire campagne entre les 2 tours. Par ailleurs, dans les des départements concernés, toujours par le scrutin majoritaire. L'embargo sur les résultats imposés jusqu'à 17h 30 est apparu tout aussi incompatibles avec la nécessité de communiquer les résultats du premier tour dès la fin de matinée et en tout état de cause avant l'ouverture du second tour de scrutin.-- Aussi même quand tu l'élection a eu a été acquise dès le 1er tour, les résultats ne pouvait pas être communiqués dans ces conditions, il n'a guère été surprenant qu'en dépit de l'embargo. Et des actions de communication mené à cette fin. Que des fuites dans les résultats étaient constaté avant 17h 30 de la part de sites Internet notamment de réseaux sociaux ainsi que d'organes de presse locale. Ainsi, la commission des lois a jugé bienvenue des aménagements. Ponctuels aux modalités de propagande et de communication. Des résultats que vise justement à apporter cette présente, proposition de loi. D'une part par la règle la dérogation de l'article L-49 du code électoral. Pour la seule période de l'entre 2 tours qui apparaît comme une mesure de bon sens. Ainsi les candidats qualifiés pour le second tour serait donc à nouveau autorisées autorisées à faire campagne, c'est-à-dire à distribuer des tracts à envoyer des messages à procéder à des appels téléphoniques en série, ou encore à à tenir des réunions électorales. Dans cette période du reste. La commission a souligné que cette disposition ne remettrait nullement en cause l'interdiction de mener des actions de propagande qui continuerait de prévaloir non seulement la veille de l'élection pour l'ensemble des départements ainsi que de toute la la journée de l'élection pour les départements concernés par le scrutin proportionnel, mais également le matin du jour de l'élection pour les départements concernés par le scrutin majoritaire. La commission a également noté que la. Dérogations visé ne remettrait pas davantage en question l'interdiction d'introduire tardivement des éléments nouveaux de polémique électorale posé par l'article L 48 2 du code électoral. D'autre part, il apparaît pertinent de rétablir la possibilité de communiquer les résultats en métropole, dès la proclamation de ses résultats et indépendamment du fait que des bureaux de vote, soit encore ouvert dans d'autres départements métropolitains, la communication des résultats pourraient ainsi s'effectuer au fil de l'eau, telle qu'elle était observé d'ailleurs avant le scrutin de 2000. Souhaité clarifier la question du remboursement des dépenses à visée électorale engagée durant la période de l'entre 2 tours par les candidats qualifiés par le second tour. La lettre actuelle de l'article L 52 tiré IV du code électoral ne permet pas en effet de considérer comme dépense électorale les dépenses qui sont engagées, le jour même de l'élection et en toute rigueur les dépenses engagées durant l'entre-2 tours des élections sénatoriales ne sont donc pas éligibles au remboursement forfaitaire de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire d'adapter la rédaction de cet article 52 tiré quatre à la spécificité du scrutin sénatorial, l'objectif étant de garantir sans ambiguïté les légitimité au remboursement des dépenses engagées entre les 2 tours de scrutin lorsque ceux-ci ont lieu le même jour, L'éligibilité aux remboursements ne signifie pas le remboursement effectif il reviendra une fine et à la Commission nationale des comptes de campagne et de financements publics de vérifier lors de l'examen de ses comptes de campagne que la dépense en question revêt bien revêt bien un caractère électoral et qu'elle s'accompagne des justificatifs requis. Voilà, mes chers collègues, le texte de la proposition de loi, telle qu'issue des travaux de la commission permettra de garantir le bon déroulement des élections sénatoriales à venir en toute logique, ce texte à vocation à entrer en vigueur avant la prochaine échéance électorale de septembre 2023 qui. Comme vous le savez verra le verront le renouvellement pardon des 170 sénateurs de la série il reviendra bien sûr au ministère de l'Intérieur d'intégrer le changement des règles hein du au futur circulaire et guide prévu à l'attention des candidats et les préfectures. Dans ces conditions, la commission des lois vous propose d'adopter la présente proposition je vous remercie de votre attention. Merci la parole est à Madame Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci. Merci madame la présidente.-- Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la proposition de loi des élections sénatoriales, porté par le président François Noël Buffet et qui a reçu un avis unanimement favorable en commission des lois. Je vais vous dire à l'aune des nouvelles fonctions combien j'attache d'importance à la qualité de nos relations service des collectivités, des territoires et de nos concitoyens. Je crois profondément au dialogue à la possibilité de s'accorder sur les meilleurs compromis et à la nécessité de dégager des consensus, je pense que cette proposition de loi qui nous a été présenté et voté à l'unanimité en commission comme je disais nous en offrent d'ores et déjà une bonne occasion. Elle porte bien sûr sur un sujet sensible car touchant à la mécanique même de notre démocratie. Mais elle se fonde aussi sur un constat que nous partageons tous, celui du caractère inadéquat des modifications de 2019 avec les particularités du scrutin sénatorial dans notre pays, notamment dans les départements concernés par le scrutin majoritaire à 2 tours. C'est pourquoi notre gouvernement porte un avis favorable sur l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi. Elles permettront de lever l'interdiction de la communication de résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, ainsi que de faire campagne entre les 2 tours des sénatoriales lorsque cela est applicable. Ce sont des mesures de bon sens qui permettent de corriger les difficultés et les ambiguïtés constatées lors de la première mise en oeuvre de ces modifications à l'occasion du scrutin de 2020. La communication des résultats dans les départements à scrutin majoritaire mais dont le 1er tour avait été conclusif avait été longuement repoussé jusqu'à la fin de la journée, alors même que les résultats fuité déjà dans les médias et par ailleurs l'impossibilité de faire campagne entre les 2 tours avait. Présenté le risque de remettre en cause la sécurité juridique des élections sénatoriales comme a pu le montrer la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel. En définitive, l'objectif qui est recherché de rendre aux élections sénatoriales. Les dispositions qui sont les plus adaptés à leurs spécificités et donc aux réalités de nos territoires pour la levée de l'interdiction de la communication de résultats, nous n'avons aucune réserve puisqu'il n'y a pas de risque de créer un précédent pour d'autres types de scrutin pour la levée de l'interdiction de faire campagne entre les 2 tours rendre inapplicable. L'article 49 du code électoral ne doit pas pour autant conduire à une politisation excessive de l'entre-deux tours afin de préserver la neutralité du vote. C'est pourquoi nous proposons simplement de reconduire les recommandations antérieures de mesure et de retenue pour les candidats au niveau infra-réglementaire comme c'était tout simplement le cas auparavant. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Je crois que ces ajustements techniques sont les bienvenus à l'horizon du prochain scrutin sénatorial et je suis convaincu qu'ils susciteront une large adhésion des sénatrices et sénateurs au-delà de tout débat passionnel. C'est une proposition de loi qui va dans le sens de l'intérêt général de notre démocratie et de la juste prise en compte des caractéristiques du Sénat chambre des territoires. Je vous remercie. Merci madame la ministre. La parole est à monsieur le président. Hervé Marseille, Marseille pour le groupe Union centriste. Et pour cinq minutes cher président.--

en matière électorale, notre haute assemblée présente toujours quelques spécificités contrairement à nos collègues députés de mode de scrutin continue de subsister pour élire les membres de notre assemblée même si au fil des réformes. Les départements soumis au scrutin majoritaire, sont de moins en moins nombreux. Des dérogations aux règles du code électoral régissant la propagande exister aussi, mais cela a assez largement disparu avec les dispositions issues de la loi Tiré 12 69 du 2 décembre 2019 qui rend applicable aux élections sénatoriales. L'ensemble des règles de propagande de droit commun jusqu'en 2014 des élections sénatoriales avait encore une autre particularité, elle n'était toujours pas soumises aux dispositions relatives aux comptes de campagne. Depuis le renouvellement de septembre 2014. Nous sommes là encore rentrer dans le droit commun. On le voit bien les particularités sénatoriales en matière électorale subsistent mais elles sont de plus en plus rares. La proposition de loi du président buffet dont je tiens à mon tour à saluer l'initiative nous invite à nous replonger dans l'organisation des élections sénatoriales. À la veille du prochain renouvellement prévu en septembre 2023. Notre rapporteur nous a précisément expliquer en quoi la loi de 2019 dont il faut rappeler qu'elle était d'initiative sénatoriale. Je rappelle que s'agissait d'une initiative. Du président Richard apportées au Sénat par notre collègue Arnaud de Belenet présenté quelques lacunes ou plutôt quelques difficultés d'application, notamment en ce qui concerne les dispositions sur la propagande entre les 2 tours pour les départements soumis au scrutin majoritaire. En effet il était peu pertinent de continuer à interdire toute propagande entre les 2 tours grâce au texte que nous nous apprêtons à voter les candidats qualifiés pour le second tour serait à nouveau autorisée à distribuer des tracts, envoyer des messages, ou encore tenir des réunions électorales entre les 2 tours. Le 2ème aspect de la PPL est un aménagement à la règle de l'embargo sur les résultats. Rappelons-nous en septembre 2020 lors du dernier renouvellement sénatorial. Nous avons vécu une séquence assez lunaire au Sénat. Presque tout le monde avait connaissance des résultats au fur et à mesure de la proclamation des candidats élus mais ici même, nous ne savions rien motus et bouche cousue jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote. Tout ceci était évidemment d'une grande hypocrisie. Avec le texte adopté en commission. Les résultats des premiers tours de scrutin pourrait ainsi être à nouveau communiqué dès la fin de la matinée, tandis que les résultats des seconds tours de scrutin et ceux des scrutins la représentation proportionnelle pourrait être à nouveau diffusé au fur et à mesure de leur remonter depuis les départements.-- Je tiens à saluer encore une fois à l'initiative du président buffet ainsi que la qualité du travail opéré par notre commission des lois sous l'égide du rapporteur notre collègue Le régulier. Il nous a permis d'ajouter en commission une utiles précisions sur le sort des dépenses engagées entre les 2 tours de scrutin en cas de journée électorale unique, autrement dit une précision sur les humilité au remboursement des dépenses liées au traditionnel déjeuner républicain d'entre deux tours pour les départements au scrutin majoritaire. Il ne faut pas exagérer quand même. l'adoption de ce texte sera de nature à sécuriser juridiquement les prochaines élections en évitant des contentieux inutile sur la propagande et les dépenses de campagne entre les 2 tours et la diffusion des résultats donc sans surprise le groupe Union centriste votera en faveur de cette proposition de loi en appelant l'attention du gouvernement. Madame la Ministre sur la nécessité d'inscrire au plus tôt ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, je vous remercie. Merci monsieur le président. La parole est à madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Il est évidemment utile à la vie des démocraties d'adapter et de corriger les règles électorales à 1 face aux difficultés ou évolution qu'elles rencontrent dans leur mise en oeuvre. Certes les ajustements techniques ne suffiront jamais pour redynamiser la culture citoyenne mais il est malgré cela impératif d'y procéder. Notre groupe salue donc l'initiative du président buffet elle participera à préserver la singularité du scrutin sénatorial. Déjà la loi du 2 décembre 2019 de notre collègue Alain Richard avait comblé quelques lacunes des règles de propagande des élections sénatoriales en prévoyant des renvois au code électoral. Ces ajustements étaient les bienvenus. Cela étant, même si je n'étais pas directement concernés. Nous avons constaté que le renouvellement de septembre 2020 s'est heurté à des limites dans l'application au scrutin sénatorial de règles de droit commun relatives à la propagande électorale il la communication des résultats. C'est limite furent au nombre de 2, elles ont été soulignée par les orateurs précédents. En 1er lieu les règles applicables en matière de propagande électorale aux autres scrutins ont été étendu aux élections des sénateurs. Cela a conduit à un ensemble d'interdiction portant sur la diffusion de tracts l'achat de publicités commerciales dans la presse ou encore la figuration de la photographie. Un second lieu l'embargo sur les résultats a été imposée jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, soit 17h 30. Celui-ci est apparu en contradiction avec la nécessité de communiquer les résultats du 1er tour de scrutin dès la fin de la mallette matinée et donc avant l'ouverture du second tour de scrutin. Au regard de ces observations. Nous sommes donc tout à fait favorable aux corrections proposées par cette proposition de loi puisqu'elles aménagent. Elles aménageur ces 2 dispositifs afin qu'ils s'accordent mieux aux spécificités du scrutin sénatorial. La commission des lois à compléter l'ensemble par des ajustements prévoyant d'adapter les règles de financement des dépenses électorales à la spécificité du scrutin sénatorial et rendant éligible au remboursement des dépenses engagées entre les 2 tours de scrutin lorsque ceux-ci ont lieu le même jour. Tout est à retenir, pourvu qu'on préserve ce qui fait la particularité du Sénat la singularité du scrutin sénatorial est l'essence même de notre chambre elle contribue à ce que nous soyons moins exposés aux fluctuations et aux arguments électoraux parfois volatile. Ce mode de désignation justifie aussi qu'en plus de participer à l'expression de la volonté générale nous assumions notre rôle constitutionnel de représentation des territoires. Tous ces mécanismes se reflète dans nos travaux, nos désaccords peuvent être profond. Ils sont toujours débattue avec sérieux la rigueur ne nous empêche pas d'être vigoureux mais toujours dans le respect de la diversité des opinions. Et pour conclure mon propos je redirai un court extrait du rapport présenté le 3 août 1874 par le député Hampton un tunnel Lefebvre Pontalis sur ce qui allait devenir la loi du 24 février 1875 instituant le Sénat de la IIIe République. Une nation et livrée à toutes les surprises à toutes les aventures car les volontés de la majorité numérique à des citoyens peuvent faire la loi. il ne faut pas que si le suffrage universel et tenté de sacrifier les intérêts de la stabilité et de la conservation nécessaires à l'existence d'une société, il puisse faire tout ce qu'il veut. Aller dans une société démocratique comme la nôtre l'importance telle est la nécessité d'un Sénat j'arrête là ma lecture mais à quelques mois du renouvellement de notre hémicycle ces quelques mots m'ont semblé pleine de justesse et pour toutes ces raisons, notre groupe votera donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. La proposition de loi déposée par le président François-Noël Buffet que nous abordons aujourd'hui permet, vous l'avez compris, d'adapter certaines dispositions du code électoral aux spécificités des élections sénatoriales le rythme régulier des consultations électorales et le signe de la vitalité démocratique et la légitimation de la représentation nationale par la désignation de ses membres au scrutin universel et la base de toute République mais la République française tient aussi sa force de l'équilibre de ses pouvoirs sous la Ve République, le bicaméralisme est au coeur de cet équilibre un parlement composé de 2 chambres différentes, complémentaires et désigné toutes les deux au scrutin universel. La particularité du mode de scrutin sénatorial. Outre d'être indirect et qu'il assure un renouvellement partiel de ses membres, gage de continuité de nos institutions. Or, lors des dernières élections de la série de du 27 septembre 2020. Certaines dispositions du code électoral sont apparus comme peu adaptées aux spécificités de la désignation des sénateurs, notamment pour ceux élus au scrutin majoritaire. 52. Circonscriptions étaient concernés en 2020. En effet, l'organisation des 2 tours de scrutin en une seule journée pour l'élection au scrutin majoritaire, n'est pas compatible avec l'interdiction de faire campagne, aussi bien la veille que le jour même. La 2ème idée inadéquation entre le code électoral en vigueur et les élections sénatoriales. Concerne l'annonce des résultats qui doivent demeurer sous embargo jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote, soit 17h 33ème inadéquation la comptabilisation des frais de campagne ne pouvant s'étendre sur la journée électorale unique comme l'a signé le président Marseille saisi natation sont liées aussi à la complexification croissante du code électoral. Ces dernières années. En 2010, la commission des Lois du Sénat avait déjà regretté la sédimentation des législations nouvelles au sein du code électoral et sa et sa perte de cohérence malgré la tentative de recodification, engagée en 2007, le chantier demeure inaboutie aussi la proposition de loi, examiné ce jour-disent à garantir le bon déroulement des prochaines élections sénatoriales en aménageant les règles de droit commun avec bon sens, la proposition de loi vise d'abord à autoriser la communication progressive des résultats dès la fin de matinée pour le premier tour et pour le second tour ainsi que ceux du scrutin à la proportionnelle pour être monté au fur et à mesure au niveau métropolitain depuis le département. Il est ensuite proposé de lever l'interdiction absurde aux candidats de faire campagne entre les 2 tours de scrutin qui ont lieu le même jour bien éloignés de la pratique notamment dans les circonscriptions concernées par le scrutin majoritaire. Dans l'optique de ces aménagements ponctuels observation pertinente été soulevée par la commission et notamment son rapporteur qui souhaite maintenir l'interdiction d'introduire tardivement des éléments nouveaux de polémique électorale qui pourrait altérer la sincérité des résultats enfin et toujours sur la proposition de notre collègue rapporteur Stéphane Le Rudulier. Et dans la logique d'aménagement proposé, la garantie de l'éligibilité au remboursement des dépenses engagées entre les 2 tours de scrutin. Dans le cas de la journée électorale unique. S'est inscrit dans la proposition de loi par souci de sécurité juridique. Si la campagne électorale pour les élections cette sénatoriale est particulière en raison du mode de désignation spécifique. Le bon déroulement du scrutin doit aussi être assurée. Force est de constater que si les élus municipaux qui remplissent pour le compte de l'État est toujours bénévolement ces formalités de vote ont un véritable savoir-faire en la matière, il n'en est pas toujours de même Madame la Ministre pour les services de l'État qui à chaque scrutin sénatorial démontre assez facilement leurs faiblesses. Or Guy à Nice la Sion Neil. Alors Madame la Ministre n'hésitez pas à transmettre aux préfectures concernées par le scrutin de 2023, un guide électoral simple et plein de bon sens pour faciliter le vote des élus locaux. Obligé de se déplacer à la préfecture et pour toutes ces raisons mon groupe votera cette proposition de loi adoptée en commission. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Alain Marc pour le groupe les indépendants et pour cinq minutes.-- Madame la présidente Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Alors que la campagne des prochaines élections sénatoriales approchent. Nous nous penchons aujourd'hui sur les conditions de ce scrutin trop mal connue par nos concitoyens mais aussi par les pouvoirs publics. Cette élection se déroule selon des modalités particulières. Le Sénat est en effet la seule assemblée élue selon deux mois de de scrutins différents majoritaire et proportionnel. Cela peut sembler étrange, mais cette différence s'explique facilement par la diversité de nos territoires. de Seine. Monsieur le président vous départements très urbanisés n'a pas grand chose à voir avec le département de l'Aveyron bien plus rural et beaucoup moins peuplée. Il est logique que tous les départements ne lisent pas leur sénateur de la même manière. En plus d'être renouvelés par moitié tous les 3 ans, le Sénat connaît les seules élections dont le 1er, le second tour ont lieu dans la même journée. Ajoutons à cela que nous sommes élus par des grands électeurs et il est clair que ce ne sera pas évident pour tous les citoyens. Ces modalités spécifiques rendent les réformes périlleuse. La loi du 2 décembre 2019 est risqué. Si le travail de notre collègue Alain Richard est à saluer, quelques difficultés sont apparues à l'usage lors du scrutin de 2020. C'est ainsi que les élections sénatoriales ont été soumises à l'interdiction de faire campagne de l'entre-deux tours. Cela peut paraître anodin mais cela quand même donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel en la matière. Un déjeuner avec des élus locaux a été assimilée à une réunion électorale avec les conséquences. Qui lui sont attachés. Si l'écart de voix étaient suffisamment importante pour que la validité du scrutin ne soit pas remise en question. Il est clair qu'une telle situation doit être sécurisé. En effet, avant la loi du 2 décembre 2019, il n'était pas interdit aux candidats qualifiés pour le second tour de faire campagne dans l'entre-deux tours. Avec la loi du président buffet il sera à nouveau possible de tenir une réunion électorale de distribuer des tracts ou encore d'appeler ou d'écrire ou grands électeurs dans l'entre-deux 2 tours. Les dépenses de campagne de l'entre-deux tours seront également éligibles au remboursement. L'autre sujet révélé par les élections de 2020. Concernant la publication des résultats.-- La loi de 2019 a imposé pour la communication des résultats de la métropole d'attendre la fermeture de l'ensemble des bureaux de vote de la métropole, bousculant les habitudes en la matière, sans que ces nouvelles règles se justifie pour ces élections particulières que sont les élections sénatoriales le dernier scrutin a donné lieu à un grand nombre de fuites sur les réseaux sociaux mais aussi par une presse accoutumés à diffuser les résultats à mesure que ceci était acquis. Le texte que nous examinons aujourd'hui propose de revenir aux règles précédentes. Permettant de publier les résultats des départements dès que ceux-ci seront connus ces dispositions emporte, me semble-t-il l'assentiment général. Les groupes de notre assemblée, s'y sont montrés favorables le gouvernement a apporté son soutien à l'adoption de ce texte lors de la procédure de législation en commission. Afin que ces quelques correctifs sont appliquées à temps pour les prochaines élections. Nous devons agir vite. Il reviendra au gouvernement d'inscrire au plus vite cette proposition à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En plus de nous permettre de mettre en lumière un scrutin trop méconnu de la plupart de nos concitoyens. Effectivement il ne, il n'y participent pas tous ce texte peut être l'occasion d'une réflexion plus profonde. Notre collègue Alain Richard a maintes fois pu attirer l'attention sur le fait que le code électoral est de moins en moins praticables en 2019 nous avons pu constater que la législation en la matière résulte d'une sédimentation de réformes et manque d'une vision d'ensemble cohérente. Il est temps d'envisager une refonte du code électoral pour donner à notre législation davantage de lisibilité et de simplicité. Je suis convaincu que cela améliorera son application diminuera le nombre de contentieux et accessoirement simplifiera la vie de tout le monde l'ensemble de notre groupe ne t'aura bien sûr en faveur de l'adoption de cette proposition de loi.

Je me réjouis vraiment. De la qualité de l'excellence de tous les orateurs qui sont intervenus avant moi, je crois qu'on a réalisé une équipe qui est vraiment une Dream Team pour cette loi. Je me réjouis, encore plus quand je vois la liste de ceux qui vont me succéder. Je pense que réellement nous allons. Faire avancer profondément en fait notre régime démocratique avec. Nos interventions et en fait nous sommes spécialiste dans l'art de la paraphrases parce que je pense que nous allons arriver à dire exactement la même chose, sans le dire, de la même façon ce qui est déjà un exploit. bon et le 2ème exploit c'est que pour la première fois je vais arriver peut-être parce que là je suis un peu lent à faire te dire d'intervention dans le temps qui parti ce qu'il y avait toujours un peu compliqué. Voilà. Donc je débarque avec. Ah bah oui y'Brest. Je ne suis pas le décompte, je comprends pas ce qu'il dit là ah voilà on repart à 0 si merci. vous connaissez le le le la position d'un coup sur l'importance des temps démocratique, et pas seulement d'ailleurs pendant les élections. Bé les élections constitue un point d'orgue les élections. Sénatoriales qui nous ont amenés sur ces bancs. On sort d'ailleurs une spécificité, il a comme particularités ce scrutin de se dérouler sur leurs 2 modalités différentes. Je pense que tout le monde l'a compris, si les orateurs été écouté selon le nombre de sièges à pourvoir l'excellent président buffet de notre commission, auteur de la présente PPL le rappeler. Dans les départements de désigner cas ou de sénateurs le scrutin majoritaire à 2 tours se déroule dans la salle et même journée. Le premier tour clos arroseur le second général ouvert dans l'après-midi dans les autres départements, il y a un scrutin de listes à la représentation proportionnelle à un seul tour. C'est ce qui nous a valu Stéphane Le Rudulier moi-même d'être élu dans les Vosges, Yonne lors des dernières élections plusieurs problèmes sont apparus dans l'application de la loi. Décembre 2019 que ce texte amende la première question c'est la possibilité officiel de utilisation de ce qu'on appelle généralement le matériel de campagne comme les bulletins de vol les mails de propagande électorale et cetera entre les 2 tours. À juste titre commission acté que cette interdiction serait contraire à la sécurité juridique des élections c'est actes Oréal sénatoriale a proposé sa levée. Cela rend possible la tenue de réunions entre deux tours la distribution de propagande. Qu'ils en fassent avec la spécificité du scrutin. Tout en rappelant le besoin de respecter l'interdiction de nouveaux éléments de polémique électorale. Les travaux de notre commission encadrer cette nouvelle propagande ressort rendant possible l'éligibilité des dépenses engagées lors de cet entre 2 tours qui peuvent être effectivement importante pour le second tour, en particulier, il faudrait quand même je pense rester un peu vigilant sur les montants des dépenses entre 2 tours qui ne doivent pas être uniquement réservée. À des agapes. Bon. 2ème problématique a été relevé lors des dernières élections, c'est la sénatoriale est Elia à la communication au public des résultats, vous l'avez dit partiel ou définitif avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Sa tête et quand je parle de métropolitains, Monsieur le Rudulier. Je ne parle pas de la métropole d'Aix-Marseille Provence. Il y a pas de polémique hein cette interdiction semble outrepasser le bon sens. Comment justifier que toujours dans le cas du scrutin à 2 tours. Les résultats du 1er tour soit proclamé mais pas publié la publicité avant le second tour, pose un problème réel et sérieux dans le déroulement du scrutin. Le présent texte décide de rectifier cette problématique et va même plus loin en permettant pour l'ensemble des scruté à sénatoriaux l'ensemble des territoires et diffusion progressive au fur et à mesure de leur augmenter par département. Voilà, chers collègues. Un texte de loi qui, quoi que très spécifique, pas d'une problématique, réelle et dans la mise en oeuvre à avoir les prochaines échéances sénatoriales de l'année prochaine permettra une consolidation de notre santé démocratique et donc, notre groupe écologiste solidarité et territoires s'associera bien entendu à une révision des règles équilibrées au plus près de la réalité du terrain.-- si Monsieur Bénard Roche je vous félicite.-- Je vais passer la parole à Monsieur Thani Mohamed Soilihi. Pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour cinq minutes.-- Madame la présidente, madame la ministre, messieurs le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Chers collègues, en mars 2019 et sur proposition de notre collègue, Alain Richard. Le Sénat avait adopté la proposition de loi visant à clarifier certaines dispositions du code électoral. Notamment celles relatives aux comptes de campagne. Plusieurs modifications était nécessaire car la sédimentation de législation nouvelle successives. Ah j'ai rendu le droit électoral peu clair voire incohérent. Pour les candidats aux différentes élections. Composée initialement de huit articles, le texte avait été enrichi et la loi promulguée en décembre 2019 contenait au final 15 articles. 15 articles éclairants qui laisse apparaître néanmoins de difficultés pour l'élection sénatoriale et qui nous concerne tous, chers collègues. Ces difficultés ont été relevées opportunément par notre président, le président du fait que je tiens à mon tour à remercier pour son initiative. Qu'ont précisé par notre rapporteur l'application. Aux élections sénatoriales des règles relatives à la propagande électorale et à la communication des résultats. En particulier dans les départements concernés par le scrutin majoritaire a montré plusieurs limites lors du dernier scrutin de septembre 2020. En effet l'interdiction de communication des résultats s'est révélé peu peu adapté aux défis aux spécificités de l'élection sénatoriale seule élections durant laquelle pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire, 2 tours de scrutin peuvent se dérouler le même jour. Ensuite les candidats qualifiés pour le second tour se sont retrouvés dans l'impossibilité de faire campagne entre les 2 tours du scrutin, conformément à l'article L-49 qui prévoit l'interdiction de mener des actions de propagande la veille et le jour de l'élection. Cette difficulté a été conforté par la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, lequel a considéré qu'un déjeuner organisé entre le 1er et le second tour de l'élection, auquel étaient conviés les grands électeurs du département devait être regardée comme une réunion électorale en prenant en compte les dispositions de l'article L-49 du code électoral. Ainsi adopté et enrichi par la commission des lois, la proposition de loi permettra aux candidats dans les départements soumis au scrutin majoritaire de faire campagne, par exemple par la tenue d'une réunion électorale entre les 2 tours de scrutin elle supprimera également l'embargo sur les résultats applicables jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de métropole. Sur proposition de notre rapporteur Stéphane Le Rudulier que je salue, pour son travail. La proposition de loi prévoira l'éligibilité au remboursement des dépenses engagées entre les 2 tours de scrutin lorsque ceux-ci ont lieu le même jour. Enfin, l'application des dispositions du texte dans les cinq collectivités régies par l'article 74 de la Constitution savoir Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon. Wallis-et-Futuna Polynésie française ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie. Ces mesures sont bienvenues. Et la fixation d'un cadre légal clair de ce que peut être une campagne entre les 2 tours vient lever toute ambiguïté, aussi le groupe RDPI votera pour cette proposition de loi. Je me permets de joindre à mon propos les rappels à de notre collègue Alain Richard sur le principe de toute campagne électorale la liberté d'expression des candidats, avec comme contrepartie, le contrôle du juge. Quant à la loyauté de l'expression des uns et des autres. Ce principe qui qui prévaut déjà appel des candidats à la prudence. Je veux souligner une règle qui sera encore plus prégnante dans la campagne de l'entre-deux tours toutes les dépenses engagées au profit d'un candidat et non pas forcément par lui-même, sont considérés comme des dépenses de campagne. Futur candidat aux candidats à un renouvellement au côté du gouvernement, nous devons collectivement rappelé ces principes de base au candidat avant l'élection. le Sénat est parfois critiqué mais nous ne voyons depuis plusieurs mois, il a un rôle essentiel de stabilisateur d'approfondissement et de contre-pouvoir si elle est l'un des grands lieux de notre République ou respect et débats apaisés sont de rigueur donnant les moyens aux futurs candidats de mener une campagne avec humilité, responsabilité valeurs républicaines dans l'espoir d'exercer ce beau mandat qui est celui des sénatrices et sénateurs de cet hémicycle.-- Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Éric Kerrouche pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes.-- Madame la présidente, madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission des lois. À ce stade de l'explication de vote, il n'y aura pas de découverte particulière, non plus, je le crains qui Guy Bénard Roche pas de demain en jouant d'être plus court que lui. Ce que je vais donc essayer de faire. Un sénateur c'est un député qui s'obstinent disait Robert de Jouvenel, hé bien je constate que notre président de la commission des Lois François-Noël Buffet montre l'inverse il est possible de ne pas s'obstiner, même quand on est sénateur et de corriger quelques défauts des textes que nous voyons se dessiner le texte que nous examinons est utile, mais il est un texte purement technique. Vous le savez, ça a été dit plusieurs fois là cette fameuse loi du 2 décembre 2019 visé à clarifier des dispositions du droit électoral singulièrement sur l'article 49 qui concerne les règles de propagande électorale. D'une part et d'autre part, s'agissant de l'article 52 de de ce même code qui concerne la. La communication des résultats électoraux, initialement, on l'a vu. Ses textes on prend origine des propositions qui ont été faites par notre collègue Alain Richard ces dispositions étaient de bon aloi. Parce que comment comprendre qu'avant cette loi, il était possible de tenir une réunion électorale le samedi mais que, en revanche pour les tracts pour les circulaires pour tout ce qui était communication électronique. Ce n'était pas possible et il était normal d'imaginer qu'il y ait une normalisation du régime de ses communications ce café ce fameux texte de décembre 2019. Il s'avère que néanmoins. Il y a des élections sénatoriales et que ces élections sénatoriales. D'ailleurs j'pour dire que à vrai dire, cette extension aux élections sénatoriales s'est fait uniquement sur amendement sans que nous les ayons alors pu mesurer l'effet concret de de ceci, il s'avère que les élections sénatoriales sont comme les élections municipales, l'une des rares élections qui connaît de mode d'élection effectivement pour. Les départements qui élisent plus de 2 sénateurs et puis un autre pour tous les autres, c'est-à-dire ceux qui sont au scrutin uninominal majoritaire. Et il s'avère qu'effectivement. La loi et dysfonctionnel singulièrement par parlant de ces élections au scrutin uninominal majoritaire et cette difficulté n'est pas qu'une difficulté théorique, elle est une difficulté pratique il y a eu un recours qui a été porté devant le Conseil constitutionnel et que la décision du 26 février 2021, montre bien que nous aurions pu avoir une annulation sur la base de cette loi de décembre 2019 et qu'il convenait dans la mesure du possible de revenir sur celle-ci alors. C'est d'autant plus vrai que nous nous préoccupons d'une élection qui arrive maintenant. Dans dans quelques mois et qu'il convenait dans la mesure encore une fois du possible de pallier l'ensemble des difficultés que nous avons pu voir d'où l'exemption de l'article L-49 du code électoral. En ce qui concerne les. Élections sénatoriales au scrutin uninominal majoritaire. Avec un ajustement qui a été trouvée par le rapporteur qui est tout aussi important, c'est très bien d'exempter. Les élections sénatoriales de l'article L-49 quand elle se déroule aussi au scrutin majoritaire, encore faut-il que les règles de financement soit également adapté et donc ces 2 dispositions. J'allais dire vont dans le bon sens. Il en va de même en ce qui concerne la communication des résultats. On a du mal à comprendre que des scrutins qui sont proclamés localement doivent attendre ensuite nationalement les séances de 17h 30. Bref. Remercier. Le président de la commission des lois pour ce texte parce qu'il vient corriger une difficulté. Technique. Demandé bien sûr au gouvernement que ce texte soit rapidement inscrit de telle façon à ce qu'ils puissent produire des effets juridiques dès les prochaines élections et puis se dire quand même que il est heureux aujourd'hui de légiférer sur ce point mais c'est ce que nous devrions faire plus. Peut être communément, c'est-à-dire tenir compte parfois du fait que la loi provoque des effets pervers et que il faut évaluer ses effets et venir les corriger, nous les corrigeons. Sur un point précis, mais le travail est grand dans tous les domaines, pour faire en sorte que justement notre Champ d'investigation aille plus loin et que nous sachions corriger les effets pervers de ce que nous votons même je vous remercie. Mais vous avez pas répondu au challenge que vous avez lancé votre collègue monsieur Bena Roche. Je vais passer la parole à Madame Cécile Cukierman. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes. Je vais essayer. Madame la présidente de le faire avec poésie. Madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord m'excuser de n'avoir pu assister au début des interventions. Pour étant retenu par ailleurs avec l'audition. Vous étiez également madame la Ministre, départ dans le cadre de la la mission de contrôle sur Lausanne. Nous. Ont également le ministre-Béchu. La proposition de loi qui. Que nous examinons aujourd'hui ne vise effectivement pas et cela a été très bien dit à l'occasion. De la législation en commission à repenser l'organisation dans dans son ensemble des élections sénatoriales ou encore de la pertinence ou non de de type de scrutin. Le même jour, selon la taille des départements et avec tout le respect que j'ai pour son auteur. Je crois qu'il ne m'en voudra pas assis j'affirme ici à cette tribune que cette proposition de loi n'a pas vocation à être révolutionnaire mais au contraire je crois à sécuriser et à améliorer le déroulement des élections sénatoriales dans les départements au scrutin uninominal puisque mais cela aussi été rappelé en l'état actuel du droit, la loi du 2 décembre 2019 à aligner le régime applicable aux élections sénatoriales en matière de campagne électorale sur celui applicable aux autres scrutins une réforme d'harmonisation qui était louable mais une extension qui a posé des difficultés. Parce qu'elle n'a pas pris. En compte la spécificité de ce scrutin sénatorial en effet durant celle-ci de tours de scrutin se déroule le même jour et de mode de scrutin s'applique d'un département à l'autre selon le nombre de sièges à pourvoir à pourvoir pour autant les candidats qualifiés pour le second tour ne sont en l'état de la loi pas autorisé à faire campagne entre les 2 tours au delà de ce que nous pourrions qualifier d'un paradoxe démocratique cette interdiction peut remettre en cause la sécurité juridique des élections sénatoriales les le démontrent les difficultés rencontrées lors des élections de septembre 2020 et la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel. La réforme des élections sénatoriales

faire campagne par exemple par la tenue d'une réunion électorale entre les 2 tours du scrutin est nécessaire. Cela répond également a besoin d'une vie démocratique riche et de la pluie, ne l'oublions pas, un entre-deux tours est un moment charnière dont nous avons tous ici fait l'expérience. Et nous pouvons convenir qu'il est tout à fait opportun de bénéficier de ce temps politique, pour le moment cloisonné ne pouvons nier qu'il s'agit de la phase ultime qui fait vivre la démocratie même s'il appartient à chacun des candidats y compris en fonction de sa personnalité en fonction de la réalité de l'histoire du département. De le faire vivre, de la manière dont il l'entend. Si donc nous rétablissons et reconnaissant par cette proposition de loi la réintroduction d'un temps de campagne entre les 2 tours, il faudra je pense continuer à travailler afin de formaliser les campagnes sénatoriales pour sécuriser les candidats mais aussi la démocratie. Nous saluons l'intégration dans les comptes de campagne des dépenses liées à ces deuxièmes tour l'égalité entre les candidats est essentielle afin que les campagnes sénatoriales soit menée de façon équitable. De plus et sur la question de supprimer Lamblin l'embargo sur les résultats applicable jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote en métropole, cela nous semble aller dans le bon sens puisque la presse locale, les sites Internet Relay déjà les résultats, bien avant 17h, il convient de noter effectivement là encore que entre les autres élections où les premiers bureaux de vote ferme à 18h et donc où le délai d'attente est de plusieurs dizaines de minutes avant 20h. Nous sommes là sur plusieurs heures et inévitablement les fuites existant autant légiférer dans ce sens. Une remarque et je veux le dire ici avec beaucoup de solennité. Si l'heure de publicité des résultats pose question comme je l'ai dit en ce que la règle du code électoral dispose que l'on doit attendent la fermeture du dernier bureau de vote en métropole pour communiquer que nous allons la modifier de fait pour la proclamation des premiers tours. Acquis des élections sénatoriales, je souhaite rappeler que toute dérogation au code électoral doit être réalisée avec parcimonie, sauf à remettre en cause les principes de ce code qui garantissent aux citoyens la sincérité du scrutin du scrutin. Mais au-delà de la confiance qui se crée. Lors de l'élection entre les électeurs et les élus au delà des différentes réserves si j'ose appeler ces remarques ainsi le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera cette proposition de loi. Qui facilite l'entre 2 tours et nous ne pouvons que souhaiter bon courage au 18 départements seront concernés par ce mode de scrutin l'an prochain. Bien merci, cher collègue. Alors je mets aux voix, la proposition de loi sur le déroulement des élections sénatoriales qui est pour. Qui est contraint qui s'abstient. La proposition de loi est adopté. Alors je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h pour le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2022. La séance est suspendue.